d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement. Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

la consommation de pesticides, ou encore celui de France Stratégie, qui propose de réformer la PAC, afin de diminuer l'utilisation d'intrants, et de procéder à un réel ajustement entre aides publiques et efforts consentis par les agriculteurs pratiquant l'agroécologie. Ce constat d'un véritable déficit d'accompagnement est ressenti par un nombre croissant d'agriculteurs, qui seraient prêts à changer leurs pratiques, mais qui se sentent insuffisamment soutenus financièrement, dans un contexte de course aux prix bas imposée par le secteur agroalimentaire et la grande distribution, mais aussi de concurrence déloyale de produits importés ne respectant pas les normes européennes et françaises.

en ce qui concerne les dotations jeunes agriculteurs, comment profiter de ce moment de renouvellement des générations pour accélérer la transition vers l'agroécologie ?

Cette décision a été bien accueillie, mais elle pose un certain nombre de questions que j'aimerais vous présenter sous la forme d'un QCM. Cela vous rappellera peut-être, monsieur le ministre, l'heureux temps de vos études de médecine sans covid. Premièrement, avez-vous réfléchi à une stratégie vaccinale pour les personnes âgées de 65 à 74 ans, sachant que la Haute Autorité de santé ne recommande pas de vacciner cette population avec le vaccin d'AstraZeneca ? Deuxièmement, la Bavière impose désormais l'usage des masques FFP2 dans les transports en commun. La plupart des scientifiques semblent penser que c'est une précaution superfétatoire. à la suite de la recommandation du Haut Conseil de la santé publique d'abandonner les masques en tissu de mauvaise qualité et de leur prohibition dans les écoles, envisagez-vous de généraliser l'interdiction des masques en tissu de catégorie 2, au profit des masques chirurgicaux Troisièmement, le Gouvernement a annoncé le déploiement prochain de tests salivaires en milieu scolaire, au retour des vacances d'hiver. Prévoyez-vous de rendre ces tests accessibles à l'ensemble de la population, notamment sous la forme d'autotests ? -ont développé des tests salivaires, validés par la Haute Autorité de santé, qui doivent être lus par un professionnel de santé. Certaines de ces start-up seraient rapidement capables de développer des autotests salivaires, qui permettraient de tester massivement la population française à domicile. Le Gouvernement est-il prêt à soutenir cette démarche française de tests salivaires et d'autotests ? Dans quelles conditions ces derniers pourraient-ils être généralisés et pris en charge par la sécurité sociale ?

dans nos écoles, de manière à pouvoir identifier, sans désagrément pour eux, des cas positifs, donc protéger et préserver l'école dont nous souhaitons qu'elle puisse rester ouverte le plus longtemps possible. Les premiers tests salivaires seront menés demain par les hôpitaux de Paris. Dès la mi-février, nous en ferons de 200 000 à 300 000 par semaine.

qui ont envie de construire- ils sont très majoritaires -, face aux objectifs actuels de la loi SRU, qui sont devenus inatteignables- tout le monde le sait ! Thierry Repentin a fait deux propositions au Gouvernement pour modifier cette loi SRU. Madame la ministre, j'aimerais savoir si le

Face à la crise que nous traversons, il est essentiel de faire mieux et de construire plus de logements sociaux. C'est l'objet de la loi SRU, qui a vingt ans cette année. Saluons la longévité et la pertinence de cette loi, ainsi que de son emblématique article 55 : plus de 1,8 million de logements ont ainsi été produits depuis 2001, dont près de 900 000 dans les communes déficitaires et soumises au rattrapage. C'est un acquis que nous pouvons tous saluer.

le Gouvernement a donné des consignes de fermeté : plus de la moitié des 550 communes n'ayant pas atteint leur objectif ont été carencées, avec parfois des reprises de permis de construire. Nous sommes attentifs à ce que les efforts se poursuivent, tout en nous mobilisant pour accompagner les communes concernées. Enfin, nous avons effectivement engagé un travail sur l'avenir de la loi SRU, dont l'échéance est prévue à la fin de 2025, ce qui conduirait à fixer en 2022 les derniers objectifs de rattrapage.

en fixant des objectifs ambitieux et atteignables et en restant fermes avec les communes qui ne jouent pas le jeu. La ministre du logement, Emmanuelle Wargon, a saisi la commission SRU, présidée par Thierry Repentin. Comme vous l'avez souligné, ce dernier a rendu un rapport et formulé des propositions en ce sens. Le rapport, rendu public la semaine dernière, fait l'objet de consultations, et ses propositions pourraient trouver une traduction législative. Peut-être aurais-je dû m'adresser au ministre de l'agriculture pour avoir une réponse un peu plus précise ... Madame la ministre, si le Gouvernement n'agit pas rapidement,

Jean-Pierre Moga, pour le groupe Union Centriste. les inondations affectent le Sud-Ouest, en particulier le département de Lot-et-Garonne. C'est une catastrophe pour les habitants.

heures, sinon vingt-quatre. Les élus ont également insisté sur le financement, l'entretien et l'aménagement des digues, difficilement supportables pour les budgets de nos petites intercommunalités.

crue. Comment assouplir les règles de curage des fossés en zone inondable afin de faciliter l'évacuation de l'eau lors de la décrue ? Des milliers de mètres cubes vont stagner des semaines dans les champs. Comment aménager les territoires et prévenir les futurs risques climatiques ?

la force cataclysmique de ces crues en énergie hydraulique exploitable ? Enfin, que répondre à nos sinistrés inquiets, qui attendent une réponse dans les meilleurs délais ? J'ai exprimé,

citoyen et écologiste. Monsieur le ministre, nous vous avions alerté sur les conséquences prévisibles de vos calculs budgétaires en matière scolaire. Eh bien, c'est pire ! Ici, ce sont des suppressions de classes au collège : celui de Blangy-sur-Bresle, par exemple, en Seine-Maritime, en perd 2 sur les 17 que compte l'établissement. Là, c'est une baisse considérable d'heures d'enseignement : au lycée de Lillebonne, par exemple, le résultat de la soustraction donne 110 heures de moins pour une réduction de seulement 22 élèves. Ce théorème vaut aussi en primaire et en maternelle, y compris en éducation prioritaire. Après avoir subi le traumatisme de deux confinements, l'éducation nationale va nous faire subir un troisième électrochoc », m'écrit le maire de Brachy, commune qui vient de réaliser un nouveau groupe scolaire. Savez-vous pourquoi cette commune a agi ainsi ? Pour répondre à vos injonctions de regrouper les écoles- injonctions qui font si mal à nos territoires ruraux et qui se voient bien mal récompensées. Une classe devrait ainsi fermer dans cette commune. Je pourrais multiplier les exemples dans toutes les académies de France. Partout, émerge la demande d'une carte scolaire qui prenne en compte la situation sanitaire et le besoin d'accompagnement renforcé des élèves, à l'image des plus de 200 élus normands qui vous lancent un appel en ce sens. La crise sanitaire n'est pas derrière nous ; les inégalités scolaires et sociales encore moins. Monsieur le ministre, allez-vous abandonner l'arithmétique de choix comptables, déconnectés de la réalité, pour faire une équation positive de la carte scolaire ?

C'est historique : plus de 500 000 contrats d'apprentissage ont été signés, soit une hausse de 40 % par rapport à 2019. Dans mon département, les Yvelines, le nombre de contrats d'apprentissage a enregistré une hausse de près de 42 passant de 6 551 à 9 311 contrats signés en l'espace de deux ans. Ces chiffres sont le reflet de la mobilisation du Gouvernement en faveur de la jeunesse. Si votre prédécesseure, Muriel Pénicaud, que je salue, a amorcé, grâce à la loi Avenir professionnel de septembre 2018, cette révolution copernicienne, en transformant le regard sur l'apprentissage et en libéralisant le système, notamment le transfert du pilotage de l'apprentissage des régions vers les branches professionnelles, vous avez, madame la ministre du travail, repris le flambeau avec brio. Vous avez su, Vous avez su, malgré la crise sanitaire, économique et sociale, maintenir et accompagner la montée en puissance de cette voie d'excellence, en instaurant, en 2020, des aides exceptionnelles allant de 5 000 à 8 000 euros, selon les situations, pour les entreprises qui embauchent un apprenti. Aujourd'hui, alors que la jeunesse est touchée par les conséquences économiques de la crise sanitaire, ce record revêt une importance cruciale. Il doit être le stimulus qui nous amènera à trouver une solution adaptée à chacun de nos jeunes pour leur garantir la même réussite et le même épanouissement que nos 500 000 apprentis. Vous l'avez dit à de nombreuses reprises, mais je le rappelle : aucun ne doit rester sur le bord de la route.

dynamique aux transformations structurelles de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, votée en 2018, qui a permis de lever les freins et de mieux adapter les formations aux besoins des entreprises. Pour maintenir cet élan dans un contexte de crise, le Gouvernement a fait le choix, dès le mois de juillet dernier, de placer l'apprentissage au coeur du plan « un jeune, une solution », avec des primes de 5 000 euros à 8 000 euros pour les entreprises. ! Les entreprises s'en sont saisies. Et ces aides se sont révélées décisives pour les TPE-PME, qui ont pu maintenir leur part prépondérante dans l'accueil des jeunes en apprentissage. Je rappelle qu'une aide de 3 000 euros est également prévue pour les collectivités locales ; je les invite à s'en saisir. Je le précise, cet élan positif a pu profiter à l'ensemble de nos territoires. Pour réussir la rentrée de 2021, une concertation s'engagera prochainement avec les partenaires sociaux, afin d'adapter les aides au contexte actuel. Mesdames, messieurs les sénateurs, notre politique en faveur de l'apprentissage est plus que jamais nécessaire. Je vous invite à la porter dans nos territoires. La parole

et je vous interrogeais sur la stratégie vaccinale du Gouvernement, tout en vous faisant des propositions. Votre réponse fut simple et limpide : « La France est prête à vacciner. » Malheureusement, les Français constatent que les choses ne

S'y ajoute l'absence de réponse à l'initiative des présidents des groupes socialistes du Sénat et de l'Assemblée nationale, Patrick Kanner et Valérie Rabault, demandant que transparence soit faite sur les contrats passés avec l'industrie pharmaceutique. Cette situation ne peut et ne doit perdurer ! Nous sommes engagés dans une course-poursuite, en France, en Europe et dans le monde, entre la vaccination et le virus, avec ses variants. Aussi, pour reprendre l'expression du Président de la République s'agissant de la guerre à mener contre le virus, nous devons mettre en place une « économie de guerre ». Monsieur le ministre, j'ai donc deux questions. Tout d'abord, allez-vous engager réellement la bataille pour obtenir la levée des licences sur les vaccins ?

d'ici à la fin du mois de février, de 2,4 millions à 4 millions de Français auront reçu une première injection. Or je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que, d'ici à la fin du mois de février, entre 3,5 millions et 4 millions de Français auront reçu une première injection. Vous pouvez le nier, mais nous atteignons nos objectifs, qui n'ont pas été revus à la baisse. Vous affirmez également que la transparence n'est pas complète concernant les contrats des laboratoires. Pour ma part, je connais le prix d'achat, le nombre de doses, les dates de livraison, le nombre de pays qui ont acheté, le prorata par rapport à la population, les dates d'achat, les dates de négociations et la nationalité des personnes qui sont allées en médiation, pour le compte de la Commission européenne, afin de contractualiser avec les laboratoires.

Depuis le 30 octobre dernier, le thermalisme est la seule offre de santé, remboursée par la sécurité sociale, qui est inaccessible à nos concitoyens. Quelque 600 000 curistes atteints de maladies chroniques, de dépression, d'obésité, accueillis dans 90 stations dédiées, ne bénéficient plus d'aucun soin thermal. Aujourd'hui, quatre mois après la fermeture des centres, les douleurs chroniques et les symptômes des curistes n'ont pas subitement disparu. Comment pouvons-nous soulager ces patients ? Devons-nous les envoyer à l'hôpital, qui est déjà surchargé ? Pouvons-nous continuer de traiter certaines affections autrement que par des médicaments parfois inefficaces ? Sur le plan économique, les établissements curistes ont réalisé 35 % de leur chiffre d'affaires en 2020, et leur trésorerie, qui affiche 110 millions d'euros de pertes, est exsangue. Malheureusement, les conséquences sont d'ores et déjà connues : des dépôts de bilan, ainsi que des mesures de sauvegarde 10 000 emplois directs non délocalisables et 100 000 emplois induits par la filière thermale sont directement menacés de disparition. En matière de développement territorial, mes collègues du groupe RDSE et moi-même vous rappelons, mes chers collègues, que 90 % des thermes sont situés dans des villes de moins de 10 000 habitants. atteint tout un écosystème, qui vacille. Ces dernières années, les villes thermales ont en effet beaucoup investi, et leurs projets de territoire marquent un véritable coup d'arrêt, faute de recettes suffisantes et prévisibles, sans compensation spécifique. Monsieur le ministre, le respect de la santé des patients est dans l'ADN de ces établissements. Des tests PCR au début de la cure, ainsi qu'en cours de cure, assortis de mesures strictes de déplacements, peuvent et doivent être mis en place. Ce protocole a fait ses preuves cet été, puisque aucun cluster n'a été constaté sur ces sites. Monsieur le ministre, dans le contexte de mal-être qui atteint tant de nos concitoyens, le thermalisme est un allié. Comment pouvez-vous permettre aux établissements thermaux, avec le concours des villes d'eau, de continuer d'assurer leurs missions de soins ? La parole

le thermalisme, comme d'ailleurs tout le secteur du tourisme, est très durement touché par la crise du covid.

le Gouvernement n'a cessé de renforcer : extension de la prise en charge de l'activité partielle aux établissements thermaux exploités sous forme de régies ; élargissement du Fonds de solidarité depuis décembre 2020, permettant l'indemnisation, sans limite d'effectifs, des entreprises ayant perdu 70 % de leur chiffre d'affaires, à hauteur de 20 % en 2019 ; mise en place d'un nouveau dispositif de compensation de 70 % des coûts fixes.

Sur proposition du secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, le Premier ministre a pris la décision de confier une mission à Jean-Yves Gouttebel, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, afin de faire des propositions structurantes pour soutenir et transformer la filière

de nouveau, un pilier du tourisme, pour que la France retrouve rapidement le premier rang des destinations mondiales en la matière. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour le groupe Les Républicains.

Sur ce secteur devait s'implanter le projet EuropaCity, sacrifié à l'automne 2019 par le Président de la République et le gouvernement de l'époque, dans un mauvais de Notre-Dame-des-Landes. Plus de dix ans de promesses, autant d'années de travail et d'investissements avaient alors été reniés, ainsi que d'importantes perspectives de développement et d'emplois pour ce territoire oublié de la République. Désolante rengaine, mais cruelle réalité malgré ce reniement lourd de conséquences pour la crédibilité de la parole publique et la confiance des investisseurs, Mme Borne avait tenu à réitérer son engagement de mener à bien « la la desserte du territoire prévue par la ligne 17 du métro du Grand Paris » et à encourager les parties prenantes à se mobiliser de nouveau pour un autre projet de développement. Pourtant, malgré cette décision prise sous l'empire d'une vision malthusienne de l'écologie, dont je déplore qu'elle ait tant infiltré l'État, les opposants n'ont pas désarmé. Au contraire, puisque, aujourd'hui, une fois encore, ils défient ouvertement l'autorité de l'État. Désormais, ils s'en prennent aux chantiers de la ligne 17 tout entière, en bloquant le puits du tunnelier. Ils prétextent un vague projet de jardinage périurbain présenté comme une solution de substitution. Ils ne voulaient pas d'un Disneyland pour consommateurs payé par le grand capital, mais ils veulent bien d'un Disneyland de la courgette pour bobos, payé par les contribuables.

en matière d'aménagement du territoire. Nous devons collectivement être en mesure d'apporter des réponses de bon sens, qui concilient le développement économique et les enjeux écologiques. Sur le fond, je puis je puis comprendre que des militants souhaitent lutter contre l'artificialisation des terres. Simplement, je pense que la méthode n'est pas la bonne et je les engage à lever ce blocage, qui pénalise l'ensemble du chantier de la ligne du Grand Paris Express, chantier dont le calendrier restera inchangé. ce qui concerne les moyens de poursuivre le développement économique et le désenclavement en matière de transport de cette zone populaire de l'est du Val-d'Oise, j'ai la conviction que l'écologie n'est en aucun cas un frein. C'est un accélérateur du développement économique,

ou une commission ! Nous n'écartons aucun scénario, y compris ceux qui permettent d'éviter d'artificialiser les rares terres agricoles de cette partie de l'Île-de-France. Bien entendu, je suis tout à fait disposée à rencontrer les parlementaires, les élus locaux, les acteurs associatifs et les citoyens du territoire, afin de définir, ensemble, les meilleures solutions pour désenclaver et développer cette partie du Val-d'Oise, qui a besoin de perspectives et de soutien. Ce n'est pas la question ! Vous aurez le soutien du Gouvernement

J'avais demandé à M. le Premier ministre de nous rassurer sur sa volonté d'expulser et j'ai entendu Mme la ministre Barbara Pompili demander gentiment aux délinquants de partir tranquillement. Je suis rassuré !

Des juges d'instruction ont été désignés, en octobre 2008, pour suivre ce dossier, après jonction des procédures initialement ouvertes aux Antilles. Ce sont les services de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, ainsi que la section de recherches de la gendarmerie de Martinique et de Guadeloupe, qui sont saisis de l'enquête sur commission rogatoire. rogatoire. Les juges d'instruction auraient signalé aux parties civiles la possible prescription de l'action publique dans ce dossier. Je le répète, nous comprenons la légitime émotion de la population et des victimes de cette terrible pollution, qui veulent obtenir, à juste titre, des réponses à leurs questions légitimes. Comme vous le savez, le Gouvernement ne peut interférer dans une procédure judiciaire en cours, ni même la commenter de quelque manière que ce soit, en vertu du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. Pour autant, il n'a cessé d'oeuvrer sur le sujet, pour les victimes, aux côtés des élus et des parlementaires. Un pas essentiel sera franchi, puisque c'est cette fois avec la participation de la société civile,

Dans la majorité des cas, les cybercriminels utilisent des logiciels, afin de crypter les données de leurs victimes, rendant inutilisable tout ou partie de leur architecture informatique. Les pirates monnaient ensuite les données volées contre le paiement d'une rançon. Particuliers, entreprises, services publics : personne n'est épargné, et les dégâts sont parfois immenses. Fait remarquable, en 2020, les attaques contre les services publics et les collectivités ont sensiblement augmenté.

Plus inquiétant encore au vu de la situation sanitaire, cette vulnérabilité n'épargne pas nos structures hospitalières, à Albertville, à Narbonne ou encore au CHU de Rouen, qui a été entièrement paralysé pendant plusieurs jours Si, fort heureusement, la santé des patients n'a pas été mise en péril, à l'avenir, des cybercriminels, plus malveillants encore, pourraient tout à fait modifier des données d'analyse médicale ou des dosages, bloquer le fonctionnement d'appareils médicaux ou chirurgicaux, ce qui entraînerait des conséquences dramatiques pour les patients hospitalisés. À l'heure où nos hôpitaux sont surchargés par l'épidémie de covid-19, un tel risque est effrayant. Madame la ministre, la vulnérabilité cyber de notre pays en fait une proie facile pour les hackers. C'est une menace de tout premier ordre. Que comptez-vous faire pour que nos entreprises et nos services publics puissent se prémunir contre ce risque ? Au-delà des actions pédagogiques, quels fonds comptez-vous mobiliser pour financer la nécessaire mise à niveau des systèmes de protection informatiques, notamment des services de santé et des collectivités territoriales ? La parole

extrêmement compétente et réputée au plan international, a été multiplié par quatre. Comme vous le savez, il existe trois types de menaces : la cybercriminalité, qui consiste à mettre la main sur des données et à demander une rançon, l'espionnage et le sabotage. Ces trois menaces doivent être prises très au sérieux, l'espionnage et le sabotage concernant plutôt les entreprises

de filière, notamment pour faire en sorte que notre offre en matière de sécurité cyber soit augmentée. Nous avons un écosystème de start-up, de grands groupes et d'universités, qui des briques de réponse face à cette menace. Elles doivent être mises ensemble pour être portées à un niveau mondial. C'est à la fois un enjeu pour les services numériques, un enjeu industriel et un enjeu pour le ministre de l'intérieur, qui est comptable

aux collectivités locales et aux structures hospitalières, pour les aider à passer un cap en termes de compétences et de matériel. Je veux donc vous rassurer : ce sujet est pris très au sérieux. Nous annoncerons la semaine prochaine

La semaine dernière, interrogée sur la rentrée de septembre 2021, Mme la secrétaire d'État Nathalie Elimas annonçait, dans cet hémicycle, un moratoire de fait pour les communes de moins de 5 000 habitants, sans l'accord du maire. Les élus locaux ont considéré ce moratoire comme acté, et je ne vous cacherai pas que la vidéo de la semaine dernière a eu un grand succès dans l'ensemble des territoires. Mais les projets de fermeture se poursuivent.

vous avez les moyens d'un moratoire ; vous avez les moyens d'augmenter le nombre d'enseignants dans les classes, devant les élèves, et c'est heureux Pourquoi ne pas dire plus clairement les choses, donner confiance et prononcer le mot « moratoire

Pour la rentrée 2020, nous avons fait une exception pour tenir compte de la crise sanitaire. Si nous le faisions année après année, nous créerions des hétérogénéités qui ne seraient pas souhaitables. En revanche, c'est vrai, il faut plus de postes pour l'école primaire. C'est la politique que nous menons. Elle permet, pour votre département comme pour tous les autres, l'amélioration

de l'insécurité dans notre pays se dégradent, et il en est un qui inquiète tout particulièrement les Français : celui qui résulte de la constitution de bandes, particulièrement dans les parties urbaines ou périurbaines de notre territoire. Le chiffre est inquiétant, puisque, au cours de l'année 2020, les agressions commises par ces bandes ont augmenté de l'ordre de 25 %, et ce sont 350 batailles qu'elles se sont livrées. Ces chiffres Ces chiffres inquiètent les Français, dans la mesure où ces bandes sont souvent constituées de mineurs, d'adolescents qui n'ont plus aucun repère moral. La violence des actes qu'ils commettent sous les caméras est là pour le démontrer. C'est aussi inquiétant parce que, on le sait, ces bandes sont en connexion avec des réseaux divers : stupéfiants, armes ou prostitution. C'est enfin terriblement inquiétant parce qu'elles savent aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux, notamment le, pour se constituer, agir et, ensuite, se dissoudre. Face à ce phénomène, il faut bien avouer que l'on ne voit pas la politique spécifique que le Gouvernement entend mener. On a même parfois le sentiment qu'il est un peu fataliste, nonchalant et passif devant l'importance du phénomène Monsieur le ministre de l'intérieur, il s'agit d'une délinquance spécifique, qui doit appeler des politiques qui le sont tout autant. Pouvez-vous aujourd'hui nous dire quelle politique spécifique vous entendez mettre en oeuvre pour lutter contre ce phénomène particulièrement inquiétant ?

Monsieur le ministre, les héros sont fatigués, car, au-delà des belles paroles, les actes ne suivent pas. Le monde rural, les agriculteurs, notamment les éleveurs, sont en grande difficulté : faiblesse des revenus, à tous, dite Égalim, lourdeur des procédures administratives, aléas climatiques, économiques et sanitaires ... Rien ne leur est épargné. Beaucoup trop d'agriculteurs vivent dans la précarité. La profession connaît un taux de mortalité par suicide très élevé. La précarité touche aussi les retraités agricoles, qui ont travaillé dur toute leur vie, 55 heures par semaine, selon vos chiffres, monsieur le ministre. Pour eux, une petite lumière se profilait au bout du tunnel avec l'adoption au mois de

pour atteindre au mieux 1 000 euros. Huit mois après le vote de cette loi, malgré les discours et les postures, les décrets d'application ne sont toujours pas parus et les retraités agricoles n'ont pas touché un centime de cette revalorisation. Pourquoi attendre, alors que cette réforme pourrait aider dès aujourd'hui de nombreux agriculteurs retraités en grande précarité ? Monsieur le ministre, la question est simple quand allez-vous signer les décrets d'application de cette loi et entériner ainsi ces avancées, même modestes, pour les retraités agricoles ?

Comme mes collègues, je rencontre régulièrement les maires de mon département. Ils nous interpellent actuellement sur d'éventuelles fermetures de classes qui interviendraient sans leur avis. Entre les inspecteurs d'académie, les recteurs, les secrétaires d'État et vous-même, les discours divergent. Monsieur le ministre, au mois de mars 2020, vous avez déclaré à la télévision vous engager à ne fermer aucune classe ni aucune école rurale sans l'accord du maire. Vous avez ajouté : « Il est très important de persévérer dans cette logique de soutien. » Interrogée ici même la semaine dernière, Mme Elimas confirmait vos propos pour la prochaine rentrée : « Aucune fermeture de classe ne s'est faite sans l'accord du maire ; il n'y a pas de raison que cela change. Ces réponses devant la représentation nationale sont sans ambiguïté : pas de fermeture de classe, d'école, sans accord du maire. Malheureusement, l'administration que vous dirigez ne l'entend pas de cette oreille ... C'est vrai ! ... et avance selon une logique exactement inverse Les cartes scolaires qui sont en cours de validation sont en opposition complète avec les engagements pris par le Gouvernement, suscitant incompréhension et colère. Les fermetures de classes mettent en difficulté les enfants, les familles, les enseignants, les maires et les directeurs Dans le contexte sanitaire actuel, au moment où les territoires ruraux connaissent un regain d'attractivité, on ne pouvait que se réjouir de l'annonce de votre décision, qui devait permettre que la rentrée 2021 se déroule dans les mêmes conditions que la rentrée 2020. Monsieur le ministre, de deux choses l'une : soit cette situation illustre la complexité, chère au Président de la République, du « en même temps », soit force est de constater que les instructions que vous donnez depuis Paris peinent à être entendues sur le terrain. Dans les deux cas, c'est votre crédibilité auprès des élus locaux qui est bousculée. Monsieur le ministre, quelle est à ce jour la réalité des engagements du Gouvernement ? Pourquoi un tel fossé entre la parole nationale et les actes sur le terrain ?

Monsieur le ministre, la suppression de classes ou de postes d'enseignants contribue au sentiment d'abandon des territoires par l'État. Les Français sont durement éprouvés par la crise sanitaire. Nous avons besoin de plus de cohérence et de stabilité dans les annonces et dans les faits pour retrouver la confiance dans la parole publique, qui est indispensable à notre démocratie

Les métros et les bus sont pleins, mais il est interdit d'aller au théâtre ou au cinéma, même en respectant le port du masque et les distances de sécurité.

De plus en plus de nos concitoyens connaissent un malaise psychologique profond. L'urgence sanitaire ne doit pas masquer l'urgence culturelle. C'est particulièrement vrai concernant nos enfants. Comment comprendre que nos écoles restent ouvertes et que, dans le même temps, les musées, les cinémas, les théâtres ou les salles de spectacle ne puissent pas recevoir de petits groupes d'élèves ? Dans ces conditions, madame la ministre, le monde de la culture ne peut plus se contenter d'espoirs vite déçus. Vous avez estimé possible la réouverture prochaine des musées et monuments.

richesse. La situation sanitaire est encore instable. Même si elle s'éclaircit relativement à certains critères, nous ne sommes pas encore complètement au clair sur les perspectives d'amélioration

avons terminé avec le débat sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion.

Les vaccins et les traitements ont permis de faire reculer les ravages provoqués par les maladies infectieuses, à tel point que l'effroi qu'elles ont causé à nos ancêtres était presque oublié. La covid-19 est venue nous rappeler les règles de base de la lutte contre les épidémies. Ces règles se résument en trois actions, qui ont connu une actualité nouvelle, mais ont aussi été reformulées à mesure que notre pays réalisait qu'il n'était pas en mesure de toutes les accomplir tester, tracer, isoler, c'est-à-dire repérer les personnes atteintes, identifier celles qu'elles sont susceptibles d'avoir contaminées, isoler les malades et les personnes contacts afin de limiter la propagation de la maladie et ainsi, progressivement, casser la dynamique des contaminations. En l'absence de vaccins et de traitements, cette stratégie est la seule disponible et elle a fait la preuve de son efficacité. Pourtant, après l'avoir consciencieusement appliquée, au tout début de l'épidémie, le Gouvernement semble y avoir tout ou partie renoncé. Les Français rapatriés de Wuhan ont été testés et mis à l'isolement dans un centre de vacances ; les personnes contaminées dans le cluster des Contamines ont été isolées à l'hôpital ; celles du cluster de Creil ont été isolées dans les conditions définies par le service de santé des armées. Mais ensuite Sur les trois pans de la stratégie, la constance, mais aussi les moyens ont fait défaut. Malgré un développement rapide, à l'honneur des équipes de recherche, les tests ont connu un déploiement hésitant et laborieux, le passage au stade industriel se révélant extrêmement complexe. Il en est résulté tout d'abord une approche malthusienne du recours aux tests, alors que certains de nos voisins testaient beaucoup plus massivement et que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) exhortait les États à le faire. Certaines capacités- les laboratoires privés, vétérinaires ou encore universitaires -ont été laissées à l'écart pour des raisons administratives qui n'étaient pourtant plus de mise dans ce Leur réintégration dans le jeu s'est faite au moment même où le revirement du Gouvernement sur l'élargissement des personnes à tester percutait de plein fouet des capacités de test encore trop peu organisées. Pendant de trop longues semaines, notre pays a testé, testé, testé, conformément aux recommandations de l'OMS, mais en pure perte, les résultats ne parvenant aux intéressés qu'une fois achevée la période où ils auraient été utiles. Pendant toute cette séquence, la détection de cas continuait à se faire à l'hôpital, pour des personnes symptomatiques, à un stade de gravité avancé et trop tard, évidemment, pour organiser un quelconque traçage. Sur le traçage, nous n'avons guère été meilleurs. La recherche d'une sophistication excessive s'est traduite par des retards et par une perte globale d'efficacité là où d'autres pays- je pense je pense en particulier à la République de Corée, dont le représentant a été entendu par la commission d'enquête -ont été mieux organisés. L'ambassadeur de France en République de Corée a insisté sur le caractère assez rustique » des moyens déployés, à rebours de l'image que d'aucuns avaient spontanément d'outils numériques qui seraient intrusifs et quasi totalitaires. Il s'agissait au contraire de mobiliser le plus de moyens humains possible et d'agir vite, ce que nous n'avons pas fait, laissant une fois de plus de côté les médecins de ville, qui voyaient pourtant dans leurs cabinets la majeure partie des personnes atteintes de la covid-19. Je serai bref, car je ne veux pas être cruel, sur l'échec, programmé d'emblée, de l'application StopCovid. Cet échec est collectif : cet outil a été conçu avec tant de prérequis que nous savions qu'il ne fonctionnerait pas. D'ailleurs, en un sens, nous ne souhaitions pas qu'il fonctionne vraiment. Cet échec a pesé sur la capacité de l'application TousAntiCovid à se faire une place dans les téléphones de nos concitoyens. Aujourd'hui encore, une majorité écrasante de cas positifs passent sous le radar du traçage, ce qui témoigne d'une efficacité très relative. Je souhaite faire une place singulière- car je sais que ma position sur le sujet n'a pas toujours été comprise -à la question de l'isolement des malades et des personnes contacts. Il se trouve que la commission des affaires sociales avait eu à se pencher sur ce sujet peu de temps avant le déclenchement de l'épidémie, à la faveur de l'examen du rapport de Martin Lévrier sur une proposition de loi de notre ancien collègue Michel Amiel. Le texte visait les cas de tuberculose résistante, mais la question est la même que faire face à un malade contagieux, qui risque de susciter une flambée épidémique ? Notre commission avait alors suggéré de donner une compétence claire au préfet. La base juridique prévue dans le code de la santé publique ayant été jugée fragile, le Gouvernement a souhaité proposer un autre cadre au Parlement. Celui qui était alors le Premier ministre avait défini ce cadre dans les termes suivants : « L'isolement doit être expliqué, consenti et accompagné. » Il s'agissait de s'en remettre au civisme de chacun : pas question d'isoler des personnes testées positives, pas question d'isoler dans les aéroports en attendant les résultats d'un test, alors même que bon nombre de nos partenaires le font, dans des conditions parfois coûteuses pour les intéressés. Des capacités hôtelières étaient pourtant disponibles pour organiser un isolement efficace, dans un contexte de mise à l'arrêt des déplacements professionnels et du tourisme. La présidente de la région Île-de-France a indiqué à la commission d'enquête avoir proposé la réservation de 7 000 lits, dont le pilotage aurait été confié à l'agence régionale de santé. C'est bien la volonté qui a fait défaut. Il peut sembler étrange, un an après le déclenchement de la crise sanitaire, de reprendre ainsi le fil des événements et de revenir sur la stratégie adoptée, alors que nous sommes toujours englués dans cette épidémie. L'objectif de la commission d'enquête était d'examiner le degré de préparation de notre pays face à l'épidémie- il est évident que nous n'étions pas prêts -, mais aussi de définir ce que nous pourrions faire pour être prêts à l'avenir. Je le répète : ce que nous pourrions faire, en l'absence de vaccins et de traitement, c'est tester, tracer, isoler. Le faisons-nous pleinement ? La réponse est « non ». En avons-nous les moyens ? Ce n'est pas certain. Le développement de tests moins contraignants reste à faire et le reste à améliorer. En avons-nous la volonté ? La question mérite d'être posée. Je vous propose de nous interroger collectivement : que ferions-nous demain devant une maladie beaucoup plus contagieuse et beaucoup plus létale pour l'ensemble de la population ? Bonne question ... Devrions-nous faire des choix et conserver la même stratégie ? J'espère que le débat de cet après-midi nous permettra de répondre à cette question. La question soulevée est tout à la fois celle de la responsabilité individuelle, de la responsabilité politique et de la confiance que les citoyens ont dans leurs dirigeants, et réciproquement. Ce n'est qu'en tirant les leçons de ce qui s'est passé que nous pourrons progresser. C'est ce à quoi la commission d'enquête s'est employée. J'espère que, sur le fondement de ses recommandations, nous pourrons avancer. La parole

permettraient à notre système de santé de tirer les leçons de cette épidémie. Ce rapport a été intitulé « Pour un nouveau départ en santé publique ».

bien -, il a beaucoup moins su construire un système de santé publique. Ce n'est pas un hasard si des pays qui ont vécu une situation épidémique en 2003 ont beaucoup mieux répondu,

On voit par exemple, dans le secteur de la culture, que persiste une réponse uniforme d'arrêt de toutes les activités, alors que vivre avec le virus en en maîtrisant au maximum la circulation pour ne pas saturer notre système de santé- telle est stratégie générale -ne nécessite pas d'arrêter uniformément toutes les activités culturelles. L'adaptation n'est toujours pas au rendez-vous, même si elle commence à être annoncée.

Le chef de l'État a annoncé que, d'ici à l'été, tous les Français qui le souhaiteraient pourraient être vaccinés. Les conditions d'un changement de stratégie vers l'éradication du virus seront-elles posées dans quelques mois ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 80 000 : c'est le nombre de victimes provisoires de cette épidémie à présent. C'est évidemment à elles que je pense au moment de prendre la parole dans cet hémicycle. Dès les premiers jours de la crise, le Sénat a agi. Il a permis au Gouvernement de prendre les mesures d'urgence qui s'imposaient. Nous avons voté, ici, en responsabilité, l'état d'urgence sanitaire et quatre Dans le but d'identifier des pistes d'amélioration des politiques publiques, la Haute Assemblée a créé une commission d'enquête dont nous débattons aujourd'hui des conclusions. Les commissions d'enquête sont d'autant plus intéressantes qu'elles cherchent à être impartiales et à faire la lumière sur des événements passés. À ce stade, nous manquons cruellement de recul pour tirer des conclusions définitives sur la gestion d'une crise à laquelle nous continuons malheureusement de faire face. La France, comme le monde entier, a subi les effets d'une pandémie qui nous a tous surpris. Certains pays, déjà habitués à ces épidémies, comme Taïwan et la Corée du Sud, ont réagi très rapidement

À l'heure où nous parlons et malgré cette opacité, les pires scénarios ont été évités. Le séquençage du virus s'est fait en quelques semaines et un vaccin a été trouvé en quelques mois. On peut, bien évidemment, regretter que la France n'en ait pas encore mis un au point- à titre personnel, je le déplore vivement -, mais le bilan -, mais le bilan que connaît notre pays pourrait être pire. Même si c'est toujours trop, la France compte aujourd'hui moins de morts par jour que l'Allemagne, pourtant si souvent citée en exemple.

Ces protections, qui ont fait cruellement défaut au printemps, sont toujours aujourd'hui l'un des piliers de notre stratégie de lutte contre la propagation du virus. Le stock de masques de l'État a été fortement asséché au cours des dernières années, celui des FFP2 a presque été réduit à néant de 2011 à 2016, celui des masques chirurgicaux a été amputé de 86 % en 2018., il apparaît évident que ces réductions ont sensiblement accru la vulnérabilité de notre pays. À en croire la tension sur le marché, nous n'étions pas les seuls à en avoir urgemment besoin. Bien sûr, d'autres ressources nous ont fait défaut, comme le curare et les respirateurs, mais ces pénuries ont été résolues plus rapidement. Au-delà de la conservation de stocks stratégiques et de la préservation de notre souveraineté, la coopération dans la résolution de la crise reste l'un des points majeurs d'amélioration. Il faudra que cette coopération soit encore renforcée entre les pays européens. l'échelon national, la coopération qui a eu lieu entre les régions en matière de santé a été positive ; nous souhaitons qu'elle se poursuive. Il convient également de permettre à la médecine de ville d'apporter tout son concours au secteur hospitalier dans ces périodes de crise, mais aussi en temps normal, pour une meilleure prévention. Il en va de même pour les capacités de test, largement évoquées par mes prédécesseurs. Il aurait été profitable d'associer les différents laboratoires, y compris vétérinaires, pour réaliser davantage de tests dans de meilleures conditions.

Enfin, il serait certainement bénéfique de mieux associer les collectivités territoriales au fonctionnement des agences régionales de santé, les ARS, mais aussi aux décisions prises par l'État. Comme souvent, nos territoires ont tenté d'apporter leur concours, mais des rigidités administratives ont freiné leurs initiatives. sont, mes chers collègues, les quelques enseignements que l'on peut tirer de la gestion française d'une pandémie qui n'est pas terminée. D'autres questions, nombreuses, restent en suspens. Elles touchent principalement à notre souveraineté économique et sanitaire, mais aussi aux conséquences de cette crise pour notre jeunesse et nos forces vives.

L'excellent travail de la commission d'enquête nous apprend que les alertes du ministère de la santé au mois de janvier ont été ignorées par l'exécutif et l'Union européenne, que le Grand Est a livré, presque seul, une bataille désespérée contre l'extension exponentielle du virus, que les choix de la direction générale de la santé, la DGS, ont empêché la reconstitution du stock stratégique de masques qui ont cruellement manqué durant plusieurs mois, information dissimulée à l'opinion par pression politique, et que ce sont les populations les plus vulnérables, les plus reléguées, qui ont été surexposées et les plus durement touchées par le virus, sans que rien soit fait alors, ni depuis, pour améliorer leurs conditions et la reconnaissance de leurs métiers. Ces manquements, ces négligences de l'État ont coûté la vie à des milliers de personnes. La responsabilité de l'État est ainsi engagée. Les recommandations proposées par le rapport sont justes. Il faut, en effet, reconstituer un stock stratégique de masques. Il faut sortir de l'hospitalo-centrisme et intégrer les établissements médico-sociaux, comme les services domiciliaires, dans notre système de santé afin de mieux protéger les populations vulnérables. Il faut faire vivre la démocratie sanitaire dans l'hôpital, mais aussi en prenant appui sur l'expertise des associations et des collectivités territoriales, proches du terrain. Toutefois, pour compléter ces recommandations et renforcer véritablement nos capacités de résilience face aux crises à venir, il semble nécessaire de rappeler également que la gravité de cette pandémie trouve aussi ses causes dans les politiques d'austérité budgétaire menées depuis des dizaines d'années, cassant l'hôpital public, déstructurant la recherche et accroissant les inégalités sociales et territoriales.

De plus, face à la pénurie de masques, de tests, de personnels, le Gouvernement n'a pas suffisamment agi, soit parce qu'il n'a pas appelé à la collaboration, soit par résistance idéologique à appliquer les lois de réquisition sanitaire. Doit être aussi questionné l'hyper-présidentialisme, qui voit se concentrer autour d'un seul un conseil de défense, un conseil scientifique, un comité d'analyse et de recherche, puis un autre conseil scientifique sur les vaccins épaulé par trois cabinets de conseil privés, qui se surajoutent à nos agences sanitaires et dont le fonctionnement reste opaque, sans contrôle public du Parlement et des acteurs du territoire. Ce chevauchement de comités et de cabinets brouille la gouvernante sanitaire et le rôle d'agences sous-dimensionnées comme Santé publique France, empêchée dans ses missions d'expertises et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Enfin, il faut que cette crise infuse une transformation profonde de nos modes de vie, car la crise découle de l'effondrement de la biodiversité. Une étude de l'université de Cambridge démontre que la migration des espèces due à la déforestation et au dérèglement climatique a permis la transmission de la covid-19 à l'être humain. Depuis vingt ans, les scientifiques nous alertent : nous sommes entrés dans le temps de la multiplication des pandémies, à la faveur de la dévastation des forêts et de la biodiversité.

La défense de la biodiversité doit accompagner la défense d'une société résiliente, respectueuse du vivant, dont le paradigme devient le soin et la justice sociale. La parole

encore inconnue il y a moins d'un an, la covid-19 a donné lieu à une crise sanitaire inédite dont l'ampleur semblait à l'époque davantage dystopique qu'envisageable. Nous sommes réunis ce jour pour un débat non sur la crise dans son ensemble, mais sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête. La constitution de celle-ci s'inscrit pleinement dans le rôle de contrôle de l'action du Gouvernement par le Parlement et relève bien de notre responsabilité vis-à-vis des Français. Cette mission est essentielle et nous y sommes évidemment favorables. Cette commission d'enquête a réalisé un travail qu'il faut souligner et que les sénateurs de notre groupe saluent : 133 personnes ont été auditionnées au cours de quarante-sept entretiens. Ces cent deux heures de travail ne permettent pourtant pas d'établir un constat exhaustif de la gestion d'une crise sanitaire mondiale aussi unique. Comment contrôler l'action du Gouvernement face à une épidémie qui faisait encore hier 439 victimes en vingt-quatre heures ? Comment critiquer des mesures sans le recul nécessaire à une analyse raisonnée et sans même pouvoir établir de comparaisons efficaces ?

de reprises, d'accalmies et maintenant de variants. Douze mois de gestes barrières à s'approprier, douze mois de vie sociale à l'arrêt. Plus de 3 millions de cas détectés et 2 millions de doses de vaccins administrées. Aussi, prenant acte des conclusions du rapport et bien que cet exercice soit indispensable, nous émettons une forte réserve quant à la temporalité de cette publication. Cette situation exceptionnelle aura forcément causé certains écueils, il serait utopique de prétendre le contraire. Pour autant, le temps du bilan arrivera, mais plus tard, lorsque les hôpitaux auront enfin un répit et que les chiffres de la contamination ne rythmeront plus nos vies. Alors, l'analyse sera efficace et essentielle, mais pas maintenant. Ce temps long nous oblige à ne pas porter de jugement trop hâtif. Ce temps long force à l'humilité. Il faut rappeler que la commission d'enquête a commencé ses travaux durant les vacances d'été, alors que les courbes étaient au plus bas. Elle les a poursuivis pendant la campagne des élections sénatoriales.

et la gestion de leurs stocks ont été le point central de bon nombre de nos discussions. Le chiffre de 1 milliard est fréquemment revenu. Les rapporteurs se sont focalisés, semble-t-il, sur un nombre sans avoir une réflexion sur la gestion exacte de ce stock. C'est pour autant bien cela qui nous a fait défaut au départ. Oui, les points d'interrogation demeurent.

Cette adaptation était cruciale, les chiffres semblent actuellement démontrer son efficacité. La ligne de crête a obligé le Gouvernement à faire preuve d'équilibre : entre liberté et restriction, entre gestes barrières et confinement, entre ouverture souhaitée de tous et fermeture nécessaire pour tous. et nous manquerions d'objectivité en affirmant le contraire, la France n'était pas prête à faire face à un phénomène totalement nouveau et d'une telle ampleur. Aucun pays ne l'était ! Pour autant, un an plus tard, le constat n'est pas aussi noir que le rapport de la commission d'enquête le souligne. Aux prémices de la crise épidémique, les évacuations sanitaires ont très largement permis de désengorger les hôpitaux des territoires les plus touchés. Je pense en particulier au territoire dont je suis l'élu. La vaccination des publics prioritaires fonctionne, la coopération européenne dont la France était moteur est établie et notre capacité de tests est exemplaire en Europe. Qui dit aujourd'hui que les tests sont gratuits en France, alors qu'ils coûtent 100 euros en Allemagne ou 300 euros au Royaume-Uni ? Le rapport Au-delà des mesures sanitaires et parce que cette crise est sociale et économique également, l'accompagnement des personnes en isolement, le soutien aux jeunes, le fonds de solidarité en faveur des entreprises et la gratuité des tests et des vaccins honorent notre pays. La solidarité dans le besoin et la fraternité devant cette situation qui touche nos citoyens de manière inégale sont les forces stabilisatrices sur cette ligne de crête que nous suivons. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, les sénateurs du groupe RDPI s'accordent à dire qu'une réelle commission de prospectives et de préconisations est importante, mais elle se fait en dehors de toute polémique politicienne et une fois la crise passée. Plutôt qu'une attitude de défiance permanente ou de critique systématique, nous préférons accompagner

collègues, dans les, Chateaubriand affirmait que « presque toujours, en politique, le résultat est contraire à la prévision ». La pandémie liée à la covid-19 était-elle prévisible ? Si, pour certains chercheurs, elle n'était pas inimaginable, son ampleur semble avoir pris le monde entier Sa gestion aurait-elle pu suivre un autre cours ? Certainement ! Peut-on en tirer des leçons sur les plans organisationnel, décisionnel et culturel ? Évidemment ! C'est ce constat qui a motivé la création d'une commission d'enquête au sein de notre assemblée. Je tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble des rapporteurs qui ont accompli un travail remarquable.

C'est dans cet esprit que je partage majoritairement les différentes préconisations de nos rapporteurs. J'axerai mon propos sur quelques points, puisque le temps qui m'est accordé ne me permettra pas de balayer les centaines de pages et l'ensemble des préconisations du rapport. Les travaux de la commission d'enquête ont tout d'abord mis en évidence l'impréparation et l'absence d'anticipation de l'État. C'est un constat largement partagé par la mission d'évaluation nommée par le Président de la République.

Corée du Sud, qui ont beaucoup appris de la pandémie du SRAS en 2003 et de la grippe A en 2009 et pour lesquels l'expérience du passé était déjà de se préparer à l'incertitude. Quoi qu'il en soit, le contexte culturel n'est pas comparable.

quasi inexistante sur notre territoire. On ne trouve plus en effet sur notre sol de véritable filière industrielle de production, la dernière usine ayant fermé ses portes en 2018.

Le premier des engagements à prendre est, bien sûr, de sécuriser la gestion de nos stocks de masques, de médicaments, de vaccins. Cela doit passer aussi par la relocalisation de leur production à l'échelle européenne.

sur la variation dans la stratégie de déploiement des centres nous a conduits à un démarrage vaccinal trop lent. Aujourd'hui, la problématique est tout autre et c'est bien : bon nombre de nos concitoyens ne peuvent pas se faire vacciner en raison d'une trop forte demande, ce qui et d'un stock limité de vaccins. Par ailleurs, certains centres sont fermés. Les rapporteurs ont également pointé une communication institutionnelle protéiforme, qui n'a pas su résister aux polémiques. Il faut reconnaître que les avis divergents, voire contradictoires, du Gouvernement et du monde scientifique ont créé de la confusion, exacerbée par les prises de position successives des experts qui ont inondé nos chaînes d'information en continu. Dans un pays caractérisé par une grande liberté d'expression, comment faire mieux ? Je l'ignore Le discours confus du démarrage a conduit nombre de nos concitoyens à déserter, dès la mi-mars, les cabinets médicaux. J'avais, à l'époque, alerté le Premier ministre et l'ARS sur les effets délétères de communiqués inadaptés qui m'étaient remontés du terrain et qui ont mis un certain temps à être corrigés. Nous n'en mesurons pas encore aujourd'hui toutes les conséquences. Enfin, cette pandémie a mis en évidence une faille dans notre mode d'organisation territorial trop centralisé, ce qui participe inexorablement à une lenteur dans la prise de décisions. C'est ainsi que les alertes émises dès le mois de février dernier par la région du Grand Est, dont je suis issue, confrontée à une vague épidémique particulièrement brutale, sont restées sans réponse. L'État n'est intervenu que plus tard, une fois que la région était dépassée. Le rapport préconise de définir les contours d'une gouvernance territoriale et d'une veille épidémiologique au plus près des réalités de terrain. C'est absolument nécessaire. Faisons davantage confiance aux élus locaux et aux personnels soignants qui ont su faire faire preuve d'une grande agilité dès lors qu'ils étaient libérés des carcans administratifs. Une transformation en profondeur est attendue

ne serait pas la dernière. C'est pourquoi j'espère que nos débats ouvriront la voie à un nouveau départ, à une année zéro de la santé publique, que les rapporteurs appellent de leurs voeux. J'ai confiance en la nature leurs voeux. J'ai confiance en la nature humaine et en sa capacité d'adaptation. Je reste optimiste quant à notre capacité collective à faire face à ce satané virus. D'ailleurs, la France, malgré les difficultés, n'est pas la plus mauvaise élève de l'Europe.

les travaux réalisés par la commission d'enquête du Sénat ont mis en lumière divers dysfonctionnements et défaillances sur la gestion de la crise de la pandémie de covid-19 et ont révélé en filigrane les raisons qui ont conduit à une telle situation. La pandémie pose en réalité une question essentielle, celle du déficit d'approvisionnement en matériel de protection, en respirateurs, en médicaments, en tests et, aujourd'hui, en vaccins Afin de répondre aux exigences de réduction du déficit public, les stocks stratégiques de médicaments, de blouses, de masques, de gants- auparavant financés par la sécurité sociale -ont été laissés à l'abandon après le transfert à l'État de la gestion des stocks de l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l'Éprus. Lorsqu'il a fallu renouveler les stocks stratégiques, l'établissement Santé publique France a été dans l'incapacité de réaliser sa mission. La logique de réduction des dépenses publiques, que nous ne cessons de dénoncer tout comme les personnels de santé et du médico-social, a montré ses limites et ses contradictions, puisque le coût du renouvellement du stock stratégique était bien inférieur aux coûts des semaines de confinement que nous avons subies. l'impréparation de votre gouvernement, les déclarations contradictoires sur l'utilité des masques, la pénurie de lits de réanimation, ne résultent pas d'un accident de parcours, mais découlent bien de choix stratégiques à l'oeuvre depuis près de trente Les conclusions du rapport sénatorial démontrent, elles, la part de responsabilité de votre gouvernement en raison de l'absence d'anticipation, de transparence et de concertation avec les soignants, les élus et les parlementaires. Le Gouvernement a perdu la confiance de nos concitoyennes et de nos concitoyens en tentant de cacher l'insuffisance des stocks de masques disponibles, puis celle des tests. Comment ne pas rappeler ici que notre commission d'enquête a par ailleurs mis de la santé est intervenu pour faire modifier un rapport d'expert sur le nombre nécessaire de masques à commander ? C'est gravissime ... Alors que l'État était aux abonnés absents, les villes, les départements, les régions, ont répondu présent et se sont mobilisés, dès le début, pour commander des masques et assurer leur acheminement auprès des populations. Ils ont continué avec la mise en place de centres de tests et aujourd'hui de vaccination. Tout cela a entraîné des dépenses considérables pour les collectivités, alors que ces financements incombaient à de l'État. En limitant les prises de décisions au cercle restreint du Président de la République autour de certains membres du Gouvernement, conseillés par un groupe d'experts et par des cabinets privés, l'isolement du pouvoir exécutif et la déconnexion avec la réalité de terrain n'ont eu de cesse de se renforcer. le Parlement- singulièrement le Sénat -à une chambre d'enregistrement, bafouant ainsi la démocratie. Des commissions d'enquête parlementaires ont tenté de rétablir la transparence et de réfléchir à l'avenir, en tirant les enseignements de la première vague de la pandémie.

il s'agit non pas de remettre en cause votre investissement personnel, monsieur le ministre, ni celui des membres de votre ministère, mais de dénoncer les choix politiques qui ont conduit à l'affaiblissement des services publics et à la déstructuration des outils de l'État. La multiplication des agences a été mise en avant comme constituant un frein à la coordination et à l'efficacité des décisions. De nombreuses auditions ont également dénoncé le nombre insuffisant de lits de réanimation, les taux d'occupation, de 90 % à 95 %, rognant toute marge de manoeuvre. Il est urgent de corriger ce manque de moyens humains, matériels et financiers dans les hôpitaux publics ; et que l'on ne nous réponde pas en citant le Ségur de la santé qui, dans les faits, n'a débouché que sur de timides revalorisations salariales, inégalitaires au demeurant, renvoyant à plus tard l'investissement indispensable dans un système de santé devant répondre aux besoins humains ! Ce n'est pas mal, tout de même ! Si telle n'est pas la première leçon à tirer de cette pandémie, alors la dégradation des conditions de travail se poursuivra, privant l'hôpital de toute attractivité, comme viennent de me le confirmer les praticiens hospitaliers, qui sont à bout et qui sont de plus en plus nombreux à envisager de partir. Gouverner, c'est prévoir. Il est urgent de répondre à l'exigence d'augmentation des capacités dans les hôpitaux, à la reconnaissance des métiers et à une révision complète de la gouvernance. La démocratie sanitaire est l'une des clefs de l'attractivité. Il faut donner du pouvoir au personnel, aux usagers et aux élus, dans des instances totalement revisitées. Une autre politique de santé est possible : renforcer les services publics et la sécurité sociale et doter les territoires de structures de proximité, comme les centres de santé, travaillant en lien avec les hôpitaux et la médecine de ville. Chaque jour qui passe démontre l'incapacité de la plupart des grands labos pharmaceutiques à organiser une production et une distribution du vaccin contre la covid-19. La France doit retrouver sa souveraineté en ce domaine. C'est tout le sens de notre proposition de création, en France et en Europe, d'un pôle public du médicament et de la recherche, qui intègre les vaccins, afin d'en faire un bien commun de l'humanité. La parole

des responsables politiques locaux, des directeurs d'hôpital, des directeurs d'ARS, des professionnels de santé, des chercheurs faisant autorité et bien d'autres encore. Le Sénat, dont la sagesse est reconnue, a présenté les conclusions de ses travaux le 8 décembre dernier. Je remercie le groupe Union Centriste et mes collègues Catherine Deroche et Bernard Jomier de m'avoir fait confiance pour être corapporteure de cette commission d'enquête. Nos critiques et recommandations ont été particulièrement pesées et je reviendrai brièvement sur certaines d'entre elles. C'est en étant lucides sur ce qui a dysfonctionné que nous pourrons avancer valablement. Le retour d'expérience sur l'année 2020 doit nous permettre de mettre en oeuvre les correctifs nécessaires, afin que notre État soit, dès à présent,

est toutefois symptomatique de ce qui n'a pas fonctionné : l'anticipation et la culture de la gestion de crise au sein du ministère de la santé. Je rappelle un fait

la suite, la gestion de celle-ci. Par ailleurs, nos auditions ont clairement mis en lumière les carences, dans les premiers temps de la crise, de la gestion centralisée. L'audition conjointe, au mois de juillet dernier, de M. Jean Rottner, président de la région Grand Est, de Mmes Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, et Brigitte Klinkert, alors présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, ainsi que de M. Christophe Lannelongue, ancien directeur de l'ARS du Grand Est fut particulièrement émouvante et révélatrice de la situation d'abandon dans laquelle s'est trouvé le territoire du Grand Est face au rouleau compresseur de Ce sont eux qui ont essuyé les plâtres et c'est de leur expérience, notamment hospitalière, que l'échelon national s'est nourri pour ensuite faire face. Il serait impensable que nous ne sachions tirer les conséquences de cette impréparation pour devenir meilleurs. Trois de nos réflexions doivent trouver un écho concret si nous ne voulons pas répéter nos erreurs. D'abord, il s'agit de renforcer le pilotage dans la réponse aux urgences sanitaires, notamment avec le rétablissement d'une fonction de délégué interministériel à la préparation et à la réponse aux urgences sanitaires (Diprus), placé auprès du Premier ministre et chargé de coordonner la vigilance permanente permanente sur l'état de préparation du pays aux crises sanitaires ou autres. Le coût humain, économique et financier de la crise actuelle doit conduire chacun d'entre nous à s'interroger sur les effets d'une politique de planification de gestion de crise court-termiste. De l'état des lieux des stocks stratégiques de produits de santé et d'équipements de protection individuelle à l'actualisation quotidienne de nos options de plans d'action, il est impératif d'assurer une veille continue de l'état de préparation du pays aux catastrophes. En effet, la crise du coronavirus aura montré et montre toujours que la réactivité des services déconcentrés de l'État

et, plus particulièrement, la notion de double tutelle, avec la responsabilité distincte des ARS pour l'aspect sanitaire et des départements pour la dimension sociale, notamment dans les Ehpad. Dans les territoires où la gestion de crise a été une réussite, nous avons constaté que le succès tenait surtout au fait que les délégations départementales des ARS et les conseils départementaux avaient su faire preuve d'initiative et d'innovation, en travaillant conjointement. Nos auditions ont par ailleurs montré combien cette coopération n'était pas naturelle. Dans les régions où les acteurs attendaient davantage les directives nationales, les difficultés engendrées par un cloisonnement trop important ont paru insurmontables au démarrage de la crise et ont fait perdre un temps précieux pour faire face à cette dernière. Les directeurs d'établissement devaient en permanence changer d'interlocuteur en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Les difficultés rencontrées dans les demandes de renforts en personnel ou l'obtention de masques en sont deux exemples. Notre rapport préconise donc une unification de la tutelle. Le fait de trancher la question de la gouvernance idéale

Enfin, si la gouvernance nationale doit être réinventée pour permettre de répondre efficacement au risque pandémique, elle doit parallèlement être accompagnée d'une refonte de la gouvernance territoriale de crise. Nous l'avons tous constaté à des degrés divers selon les territoires, la relation entre préfets et services des ARS a, pour le moins, manqué de fluidité. Dans le département du Jura, de l'ARS a fait beaucoup et bien avec très peu de moyens. Toutefois, notre action gagnerait en efficacité en réaffirmant un simple fait : la gestion de crise, c'est l'affaire du ministère de l'intérieur. Nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion sur la clarification du pilotage territorial de crise sanitaire, car ce sont les échelons déconcentrés qui, avec les collectivités locales, répondent, aujourd'hui encore, à la crise. Leur préparation, les procédures à appliquer pour travailler conjointement sont des questions centrales. La campagne de vaccination est un exemple très actuel de ce besoin d'anticipation. Là encore, les préfets, les délégués territoriaux d'ARS, les maires, les présidents de collectivités territoriales doivent s'adapter et composer, du jour au lendemain, pour réparer les erreurs qui auraient pu être évitées. Depuis plus d'un an, ils sont systématiquement dans l'urgence. premier trimestre 2020 est loin derrière nous. Puisque notre monde a changé, puisque nos vies changent, il faut accepter de changer l'État. La

Le constat a été dressé par les intéressés eux-mêmes : il est nécessaire de renforcer la fluidité des relations entre les préfets et les directeurs généraux des agences régionales de santé. Cette question est déterminante pour les élus locaux, plus familiers d'une relation étroite avec le préfet de département qu'avec le directeur général de l'ARS. En temps de crise, l'organisation de cette relation est clairement prévue par le code de la santé publique : le préfet peut prendre les commandes. Ce texte existe et il n'est pas nécessaire d'en inventer un nouveau. Pourtant, il n'a pas été utilisé, ce qui nous donne à penser que le défaut d'organisation était plus général et pas seulement lié à l'existence même des ARS. C'est pourquoi la commission d'enquête du Sénat, à la différence de celle de l'Assemblée nationale, n'a pas préconisé leur suppression. nous avons souhaité que des redéploiements interviennent au sein des ARS, afin de permettre d'armer correctement les délégations départementales, qui ont trop souvent semblé dépourvues d'informations, de moyens et de capacités de décision. la réforme des régions a percuté celle des ARS, dont les sièges sont souvent trop éloignés du terrain. Nous pensons que le délégué départemental de l'ARS doit prendre des responsabilités dans la gestion des crises, en déclinant, dans son département, un plan pandémie et en disposant des données épidémiologiques nécessaires, les cellules d'intervention en région de Santé publique France étant elles-mêmes intégrées au sein des ARS. Ces données épidémiologiques devraient également permettre d'apporter des réponses différenciées à des territoires placés dans des situations différentes. Le cas emblématique de la première phase a sans doute été celui de la Guyane, entrée en confinement alors que sa situation ne le justifiait pas forcément et privée de cette mesure en pleine flambée de l'épidémie. Le pilotage de la crise s'est alors clairement révélé comme trop centralisé et il ne semble pas que ce point ait significativement évolué dans la durée. En matière de recherche, l'effort a été tout à fait exceptionnel et les résultats ont été au-delà des attentes que nous pouvions avoir. Le développement des vaccins en est un exemple. En France, pourtant, cet effort de recherche a paru trop dispersé et, de fait, il a conduit à des résultats limités.

Il nous semble qu'une démarche similaire aurait pu être conduite en France ; les ministères chargés de la santé et de la recherche doivent pouvoir, selon nous, assurer la définition de travaux prioritaires, qui pourraient concentrer les financements exceptionnels mobilisés pendant une crise.

sur la méthodologie en matière de recherche clinique, laissant se déclencher sur la place publique des controverses, qui n'ont fait qu'alimenter le désarroi et la défiance de nos concitoyens. Il nous a également semblé que la recherche sur les maladies émergentes et infectieuses gagnerait à mieux se structurer. C'était l'objet du consortium REACTing, qui n'a pu assurer cette mission Pourrez-vous préciser, monsieur le ministre, les missions et les moyens de la nouvelle agence, fondée sur REACTing, dont vous avez annoncé la création ? Pour sa part, la commission d'enquête a recommandé la création d'une structure dédiée à la recherche en maladies infectieuses, en rapprochant le consortium REACTing de l'Agence nationale de la recherche sur le sida et les maladies infectieuses, dont la mission est de fédérer, coordonner, animer et financer toute la recherche publique sur le sida et les hépatites virales. Cette capacité à fédérer a clairement fait défaut dans la recherche contre la covid. D'une façon plus générale, quels enseignements le Gouvernement tire-t-il de cette crise en matière de recherche ? Tout comme l'hôpital, le secteur de la recherche était en crise et en proie au doute bien avant le déclenchement de l'épidémie de covid.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'épidémie est encore là ; elle nous oblige à la plus grande vigilance, tant dans notre vie quotidienne que dans les analyses et les jugements portés, lesquels ne sauraient être définitifs. L'heure n'est pas encore au bilan, même s'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour tenir un débat démocratique. Voilà un an, le virus était encore très largement un mystère à percer, une menace abstraite, un risque mal défini. Aujourd'hui, c'est un ennemi mieux identifié, qui a sévi partout dans le monde- j'y insiste provoquant plus de 80 000 morts dans notre pays. Nous faisons donc face à une épidémie évolutive, que nous suivons chaque jour, heure par heure, sur laquelle les connaissances, elles aussi, évoluent sans cesse, tout comme évoluent les outils qui nous permettent de lutter, avec toujours plus d'efficacité, contre ce virus. Je salue une nouvelle fois tous ceux qui se mobilisent depuis de longs mois, sans compter leur temps ni leur énergie. Tout notre système de santé a été mis en tension, comme jamais auparavant ; toutes les structures économiques et sociales de notre pays ont été bouleversées ; tous les Français ont dû apprendre à vivre autrement, pour éviter le pire. Il a été question de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne. Ce qui est sûr, c'est que nous vivons une épreuve collective majeure, une épreuve inconnue de notre génération- de la mienne, de la vôtre -, une épreuve qui n'épargne personne et qui demande à chacun des efforts et même des sacrifices. Une crise, c'est une perte de contrôle, c'est un événement qui surgit, qui prend de court, qui nous dépasse d'abord et auquel nous nous adaptons ensuite. Aujourd'hui, nous avons davantage de solutions pour combattre l'épidémie et nous avons repris sur elle un contrôle relatif. La vaccination est un espoir formidable, un outil aussi puissant qu'inespéré il y a encore quelques semaines. Toutefois, mesdames, messieurs les sénateurs, des variants apparaissent déjà, qui se développent aux quatre coins du monde, qui posent de nouvelles questions, de nouvelles difficultés, de nouveaux défis et qui peuvent mettre à mal notre stratégie.

À ce jour, à l'heure même où nous parlons, nous disposons de temps intermédiaires, mais la ligne d'arrivée n'a pas été franchie. Le travail d'analyse doit impérativement tenir compte de cette donnée. Pour autant, ce travail est indispensable et nous devons préparer ensemble notre système de santé pour demain. On appelle cela « tirer les enseignements » ; c'est notre responsabilité. Des engagements forts ont déjà été pris, par exemple avec le Ségur de la santé, qui répondait à des revendications anciennes et légitimes formulées par les soignants. Nous avons revalorisé, dans des proportions inédites, les métiers du soin ; nous avons investi comme jamais, pour donner à l'hôpital public les moyens d'affronter tant le quotidien que des épreuves de grande ampleur. Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis engagé dans la gestion de cette crise sanitaire depuis la première minute de ma prise de fonction. Dans quelques jours, cela fera un an que j'ai été nommé ministre des solidarités et de la santé. Par temps calme, ce ministère n'est pas comme les autres, puisqu'il touche à ce que chacun a de plus précieux : sa santé et celle de ses proches. Dans la tempête, ce ministère cristallise les attentes, les espoirs, les angoisses de tout un pays. En franchissant les portes du ministère, je savais que ma responsabilité serait immense et, chaque jour, j'ai mesuré ces attentes, ces espoirs et ces angoisses. Je n'ai pas commenté en différé. J'ai agi en temps réel et l'intérêt général a été ma seule boussole. Nous allons

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

si la réponse à l'urgence peut, par essence, être imparfaite, des leçons durables auraient dû être tirées de la crise. Les choix politiques, les égarements stratégiques n'ont pas été assumés ; nous le regrettons. L'ampleur du choc ressenti par notre pays depuis bientôt un an est inédite. Nous faisons face à un bilan humain sans précédent et à une urgence sanitaire et sociale. Le début de crise a été marqué par un manque d'anticipation, une absence de prise de décision et une accumulation des dénis. La première défiance est la vôtre, monsieur le ministre, c'est une défiance à l'égard des Français, pointés du doigt comme de mauvais élèves peu respectueux des consignes, accusés d'emblée d'être de potentiels vecteurs de la maladie au comportement insouciant. Ce qui en résulte en retour- principe de réaction -, c'est de la défiance, accentuée par l'incompréhension de vos mesures.

par le truchement du conseil de défense. Aujourd'hui, elle accuse le coup de sa verticalité : notre démocratie a été mise à mal. La stratégie des masques, des tests et des vaccins n'a clairement pas été à la hauteur. Nous avons l'impression persistante d'être toujours en retard. Ma question porte sur l'expertise et sur le rôle du conseil scientifique mis en place à la hâte. N'aurait-on pas dû avoir d'entrée de jeu une instance autonome, pérenne, multidisciplinaire, indépendante, dotée de moyens importants et capable de faire face aux crises à venir, dépassant le strict champ des pandémies,

Madame la sénatrice, on pourrait disserter longtemps pour savoir si une crise s'anticipe. Par définition, si une crise est anticipée, il y a moins de risques qu'elle survienne ... La crise a éclaté en France, dans toute l'Europe, dans le monde entier. On peut donc considérer qu'il y a peut-être un facteur qui échappe aux politiques publiques et aux particularités

Le même constat a été dressé en ce qui concerne la vaccination et les tests de dépistage, qui n'ont pu se faire de façon massive que grâce à l'intervention des collectivités locales. Le manque d'anticipation constaté, les difficultés logistiques, l'absence de prise en compte du secteur de ville, ont mis en évidence la nécessité d'une territorialisation de la prise en charge sanitaire de nos concitoyens. Cette territorialisation est attendue de tous- élus et professionnels de santé -dans nos territoires.

Quant aux quelques CPTS existantes, elles n'auraient pas été sollicitées dans la gestion de la crise et ne le sont toujours pas pour la vaccination anti-covid. Pourtant, les CPTS pourraient contribuer à une organisation fine du « dernier kilomètre ». Elles pourraient également permettre la déclinaison, à l'échelon local, d'un plan pandémie coordonné avec les élus des collectivités territoriales, sous la responsabilité du délégué départemental de l'ARS, comme cela est suggéré dans le rapport.

très rapide des CPTS dans les territoires ; vous en avez parlé et vous avez raison : partout où elles se trouvent, ces communautés font l'unanimité des soignants, des usagers et des élus, fait suffisamment rare pour être souligné.

que les liens entre les ordres médicaux, les syndicats médicaux, les représentants du monde hospitalier et les élus locaux se sont renforcés. Par exemple, pour la vaccination, dans tous les départements se trouvent des comités de pilotage départementaux. Je m'entretiens régulièrement avec un certain nombre d'entre eux, j'étais ainsi virtuellement avec celui

a causé la mort de nombreux Français. J'ai une pensée pour eux et pour leurs proches. Malgré les difficultés, notre système hospitalier a tenu bon grâce au dévouement de nos soignants, auxquels je veux rendre hommage. L'ensemble des services de l'État, tout comme les collectivités territoriales, sont mobilisés depuis le début de cette pandémie afin de protéger au mieux nos concitoyens. Face à un virus inconnu et mutant, la tâche est loin d'être simple. Nos territoires n'ont pas été touchés par la maladie en même temps ni avec la même intensité. Les ARS n'auront donc pas été confrontées aux mêmes réalités. De nombreux élus locaux ont eu le sentiment que ces agences n'étaient pas suffisamment proches du terrain. De manière plus générale, un sentiment de déconnexion de l'administration a été partagé, notamment par ceux qui ont à appliquer des protocoles sanitaires destinés aux établissements recevant du public, comme les écoles ou les commerces. Ces documents ont fait l'objet de nombreuses modifications et se révèlent parfois trop éloignés des réalités matérielles pour être applicables. Une association plus étroite des collectivités aurait pu sans doute lever quelques difficultés. Aussi, monsieur le ministre, ma question est simple : pensez-vous que rapprocher l'administration du terrain et mieux associer les élus locaux à l'action des services de l'État soit nécessaire et utile ? Comment comptez-vous procéder concrètement pour améliorer la situation ? La parole

En prenant quelques instants pour regarder comment nos voisins gèrent la pandémie depuis un an, on constate rapidement qu'aucune démocratie ne fonctionne avec une aussi grande verticalité que la nôtre. Ce qui était acceptable il y a un an est devenu insupportable aujourd'hui. Je rappelle brièvement que, après être allé au théâtre pour rassurer les Français au début du mois de mars dernier, le Président de la République a décidé, huit jours plus tard, sans aucun cadre légal, de confiner le pays. Nous ne lui tenons pas rigueur d'une décision qui s'imposait et que nous avons d'ailleurs validée, mais je mobilise cet exemple pour préciser que notre politique de gestion de crise ne peut plus relever du seul chef de l'État. L'exemple du confinement avorté, qui, voilà quinze jours, a pris par surprise jusqu'au Premier ministre, est une nouvelle illustration de cette situation délétère. Ce manque de visibilité est aussi pesant et usant pour nos concitoyens que les mesures de restriction de liberté. liberté. Que faire face à cette crise, qui est, hélas, partie pour durer ? Il me semble que l'Afrique du Sud, pays pourtant très durement touché par le virus, a pris le temps d'élaborer un mode de gouvernance intéressant

de la liberté de mouvement et d'activités. Le changement de niveau est activé par le gouvernement sur la base de critères objectifs : circulation du virus, nombre de décès, niveau d'occupation des hôpitaux, avec, bien sûr, une possibilité de territorialisation. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui empêche le Gouvernement de travailler sur un dispositif semblable et, en tout cas, de travailler sur le temps long et sur l'adaptation dont vous avez parlé ? Cela permettrait de donner de la visibilité aux Français et aux Françaises, aux élus locaux et aux entreprises et, surtout, de renforcer l'acceptabilité des mesures et de soulager notre démocratie.

C'est dans l'esprit des chartes de confiance en matière d'événements sanitaires indésirables qu'il convient de tirer certaines leçons de la pandémie de covid-19. Nous ne demandons pas de prévoir l'imprévisible, car nous ne souhaitons pas une vie sans imprévu. En revanche, il convient que la société soit agile et réactive face à toute situation inattendue et que nous soyons dotés de la capacité de répondre aux crises, surtout lorsque celles-ci touchent l'ensemble de la population. La résolution d'une crise, ce n'est pas le retour en arrière. Ce n'est pas non plus une révolution : on sait très bien que, après avoir viré à 360 degrés, on se retrouve généralement à la même place ... Ce doit être le départ d'une nouvelle organisation, qui tire les conséquences de cette crise : après ne sera plus comme avant. La santé est un tout. Le bien-être physique, psychique et social des individus nécessite une parfaite harmonie entre le médico-social et le sanitaire. Les doubles tutelles sont un handicap pour cette harmonie. Monsieur le ministre, en tirerez-vous les leçons pour rassembler ces compétences ? Il en est de même des relations entre ARS et préfet. Comptez-vous unifier l'autorité de l'État pour éviter les atermoiements en cas de crise ? Nous avons également mesuré l'implication des collectivités dans les réponses apportées.

Enfin, trop de communication tue la communication. Il serait tellement plus clair de savoir quelle est la seule autorité scientifique ayant légitimité à s'exprimer, afin que la communication du Gouvernement se fasse dans la clarté et la transparence, comme je vous l'ai déjà demandé pour la stratégie vaccinale.

Certains, en responsabilité, ont une expression qui est à la fois mesurée, ordonnée et conforme aux données de la science, d'autres non, mais notre État ne censure pas ses scientifiques et ses médecins.

Le ministère de l'intérieur sait gérer des crises qui sont propres à la sécurité publique. L'armée est à même de gérer un certain nombre de crises qui relèvent aussi des missions régaliennes. La question de logistique, y compris du secteur privé, relève de la compétence de tout l'État- on me le reproche suffisamment.

aurait pu anticiper la deuxième vague de covid-19 bien plus tôt. Malheureusement, monsieur le ministre, vous n'avez pas écouté les mises en garde. Surtout, vous n'avez pas tiré les leçons des échecs de la gestion de la pandémie au premier trimestre 2020. Face à la crise, des solutions alternatives ont émergé des territoires. Les élus se sont mobilisés pour la fabrication de masques. Je pense également aux initiatives de fabrication de masques lavables au sein de la filière textile. La commission d'enquête sénatoriale préconise d'ailleurs de promouvoir ces masques produits en France et de pérenniser la filière. La mise à disposition d'une production nationale de masques grand public mobilisables rapidement en cas de crise sanitaire est aujourd'hui nécessaire. Monsieur le ministre, depuis lundi, l'usage des masques artisanaux est interdit à l'école et les masques de catégorie 1 sont obligatoires. Actuellement, aucune homologation n'est prévue pour la commercialisation des masques. Que prévoit le Gouvernement pour aider les initiatives locales de production de masques de la filière textile à obtenir la certification de catégorie 1 afin de maintenir cette activité sur notre territoire ? Enfin, monsieur le ministre, nous vous proposons d'envoyer à chaque enfant scolarisé des masques de catégorie 1, par le biais des communes ou des communautés d'agglomération. Qu'en pensez-vous ? à vous remercier

puisque nous avons réalisé le troisième envoi de 45 millions de masques gratuits à 7 millions de Français précaires et le troisième déstockage de plusieurs dizaines de millions de masques à usage unique à destination des personnes qui vivent

savoir si vous êtes d'accord ou non avec cette proposition de fournir à tous les enfants scolarisés un masque, qu'il soit dans une famille où l'on gagne le SMIC ou dans une famille

La pandémie que nous traversons a eu la vertu de révéler, dans certains cas, les faiblesses de la gouvernance territoriale de crise. Les conclusions de la commission d'enquête, dont je salue la finesse et la clarté, le confirment : en matière de santé, la décentralisation est insuffisante et la déconcentration reste maladroite. maladroite. La décentralisation est insuffisante. Le pilotage de la gestion de crise est apparu trop centralisé. Concrètement, les collectivités territoriales n'ont pas été suffisamment associées aux décisions. Or elles sont des sismographes indispensables pour enregistrer les signaux faibles et les spécificités de nos territoires. Elles seules peuvent garantir un calibrage fin d'une politique de santé publique. En effet, les cibles d'une telle politique ne sont pas hors sol. Elles sont charnelles : ce sont des femmes et des hommes qui habitent des communes, des départements, des régions. En matière de santé, la déconcentration est maladroite. Comme le soulignent les conclusions de la commission d'enquête, les agences régionales de santé, services déconcentrés de l'État, ont pratiqué une gestion de crise trop éloignée du terrain. Leur délégation départementale n'a pas pu jouer un rôle d'interface efficace avec les élus locaux.

comment comptez-vous les rendre possibles ? Seriez-vous d'accord pour recentrer les missions des ARS autour de l'organisation et de la coordination de la politique de sécurité sanitaire, de santé publique et de santé au travail, régionaliser la convention d'objectifs et de gestion signée tous les cinq ans entre l'État et la Caisse mettre en place une double expérimentation de déconcentration et de décentralisation accrues en matière de santé dans les régions volontaires, en transférant les compétences des ARS aux régions Ces questions sont complexes, mais se veulent constructives. Nous restons par ailleurs attentifs au principe d'égalité de traitement, qu'une décentralisation ne doit pas menacer. La parole

a été ressenti chez les personnes malades et en situation de handicap ainsi que chez leurs proches aidants, parfois amenés à gérer des soins curatifs et palliatifs.

Ils ont fait de leur mieux. Il est donc nécessaire de mettre fin à la centralisation excessive du pilotage opérationnel des instances de santé, en mettant en avant les complémentarités et potentialités des différents territoires.

Enfin, monsieur le ministre, comment comptez-vous valoriser les différentes instances de démocratie sanitaire concernées dans la proximité et la démocratie ? La parole est à M. le ministre. Madame la sénatrice, j'ai participé lundi aux travaux du conseil départemental d'analyse et de vigilance du Gers, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette initiative locale peut servir d'exemple. Elle est promue par le président du département, Philippe Martin, que vous connaissez bien. Elle travaille main dans la main avec l'État et ses services. Elle réunit les professionnels de santé et des citoyens

dont je rappelle que le Président de la République l'a qualifiée de « temps de guerre ». Cette gestion de crise n'a manifestement pas permis d'assurer une territorialisation dynamique des décisions qui aurait

crise. À cette époque, loin d'être linéaire, la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre le covid-19 s'est plutôt apparentée à une course d'obstacles. Il a fallu

aujourd'hui remédier à cette gestion lente et désordonnée de la crise sanitaire, qui participe d'une certaine manière au climat anxiogène ressenti par les Français ?

le ministre, pendant deux mois, la direction générale de la santé (DGS) enjoignait chaque soir les Français de faire preuve de responsabilité face au covid-19. Aujourd'hui, nos concitoyens sont en droit de demander à l'administration de faire preuve de la même responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité ? C'est l'obligation de répondre de ses actes et, le cas échéant, de ses fautes. Je me concentrerai ici sur quelques-unes de celles qui ont été commises par la DGS. La lecture de notre rapport permet d'identifier trois fautes majeures. La dissimulation, d'abord : mise au courant dès 2018 de la non-conformité et du caractère périssable de centaines de millions de masques, la DGS n'en informait sciemment pas la ministre de la santé. L'impréparation, ensuite : la DGS décidait de ne pas reconstituer ce stock, toujours sans en informer le Gouvernement et, par là même, les Français. La manipulation, enfin la pénurie arrivée, la DGS faisait pression pour modifier un avis scientifique sur la nécessité de disposer d'un stock élevé de masques. Dissimulation, impréparation, manipulation : trois fautes majeures, aucune responsabilité,

Monsieur le sénateur, je ne crois pas être devant une cour de justice à devoir répondre d'accusations au nom de mon directeur général de la santé. J'ai déjà eu à m'exprimer sur cette question. J'ai lu le rapport de la commission d'enquête ; les éléments qui y figurent ont été envoyés par le directeur général de la santé lui-même. J'ai eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises qu'il avait toute ma confiance et je le remercie de l'action qu'il mène au service de l'intérêt général. Ce n'est

depuis un an : notre pays n'était pas suffisamment préparé à la gestion d'une telle crise sanitaire. Nos sphères décisionnelles et scientifiques étaient mal coordonnées et la communication de votre gouvernement n'a pas toujours su convaincre du bien-fondé de certaines dispositions, Les mois ont passé et une recherche assidue sur de futurs vaccins a porté ses fruits. Depuis le mois de décembre dernier, plusieurs vaccins sont autorisés et leur injection selon une stratégie établie par la Haute Autorité de santé (HAS). Cet aboutissement d'intenses recherches et de découvertes antérieures innovantes a suscité beaucoup d'espoir. Pourtant, la coordination opérationnelle pour le déploiement de la vaccination chez les publics prioritaires a connu quelques déboires au début du mois de janvier dernier : sans l'appui logistique des collectivités, ni les ARS ni les préfectures n'étaient capables de déployer les centres de vaccination. Nous avons de nouveau fait face à un manque d'anticipation en haut lieu que le tirage au sort d'un comité citoyen a vainement tenté de dissimuler. À ce jour, les mêmes griefs persistent : pour l'injection du faible contingent de doses disponibles, les files d'attente sont gérées au jour le jour, quelques créneaux libérés ici et des annulations massives là. Il a fallu attendre un mois de campagne vaccinale pour que les données opérationnelles de date de livraison et de niveau de stocks soient rendues publiques. Désormais se pose la question de l'adaptation de notre stratégie vaccinale à l'apparition des nouveaux variants. Ma question est simple : combien de semaines faudra-t-il encore attendre pour disposer d'une information mise à jour et éclairée sur l'adaptation de notre stratégie vaccinale et sa déclinaison territoriale face à la circulation croissante des nouveaux variants ? La parole Madame la sénatrice, les informations sur une évolution éventuelle de la stratégie vaccinale arriveront quand nous les aurons, c'est-à-dire quand nous saurons si les vaccins sont efficaces sur tel ou tel variant, quel vaccin il faut pour quelle personne et quand ces éléments seront validés par les autorités scientifiques

pour définir les politiques de lutte contre les pandémies, mais il aurait surtout intérêt à le faire pour décliner ses politiques territorialement et localement. Il y a une évidence : les décisions que prend l'État qui créent un certain nombre de difficultés et de l'insatisfaction provoquent des plaintes qui sont adressées en priorité aux collectivités territoriales. Monsieur le ministre, comment entendez-vous

Monsieur le ministre,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on a beaucoup évoqué la mémoire de Louis Pasteur ces derniers temps. À l'heure où les vaccins sont au centre de toutes les attentions, ce bienfaiteur de l'humanité, gloire de la III République et fierté française, méritait bien ces hommages. On a moins parlé de René Descartes. À juste titre, car, au coeur du tourbillon de contradictions qui souffle sur notre pays depuis un an, ce chantre de la raison, incarnation de la déduction logique, serait bien en peine de s'y retrouver. La boussole de la parole publique est devenue baroque. Lundi, l'Élysée dit « rouge » ; mardi, Matignon affirme « bleu » ; mercredi, Ségur nuance « vert Trois exemples suffiront à illustrer ce qui n'est malheureusement pas une caricature. D'abord « faussement protecteur », le masque est devenu « salvateur » et son oubli a valu des dizaines de milliers de verbalisations à un tarif sévère. Tolérance zéro pour deux clients dans un restaurant, mais feu vert pour cent adolescents dans la cantine d'un collège, ainsi que pour quelques ouvriers du bâtiment dans quelques auberges chanceuses. Au mois de novembre dernier, on ferme les petits commerces non alimentaires en laissant ouvertes les grandes surfaces. Aujourd'hui, on ferme les grandes surfaces et on laisse ouverts les petits magasins. Comprenne qui pourra ! « Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis » semble être la devise du Gouvernement. Pas sûr, toutefois, que les 66 millions de Français, qui ne sont ni des béni-oui-oui ni des procureurs, apprécient. Un peu de bon sens- « la chose au monde la mieux partagée », selon Descartes -n'a jamais nui. Permettez-moi, pour terminer, une suggestion, qui ne porte pas sur la territorialisation, car il en a beaucoup été question, mais concerne plusieurs centaines de milliers de jeunes. Notre hémicycle n'est-il pas comparable à la plupart des amphithéâtres d'université, aujourd'hui désertés, au grand dam des étudiants, qui supportent de plus en plus mal l'isolement auquel on les condamne ? Ne pourrait-on pas permettre aux étudiants ce que l'on autorise aux sénateurs et députés, ... Allons bon ! ... à savoir se réunir à demi-effectif ? Doit-on considérer nos jeunes comme irresponsables et incapables de respecter un minimum de précautions sanitaires ?

Cinq, on a permis à un contingent d'étudiants de commencer à revenir dans les universités, en faisant attention à ce qu'ils ne soient pas très nombreux. Je note, monsieur le sénateur, sans vouloir vous taquiner, que l'on est ici très loin ici d'un amphithéâtre bondé d'étudiants ...

Face à ces constats, la commission d'enquête a formulé un certain nombre de propositions. Comme nous le savons tous, la crise sanitaire a touché de plein fouet les plus vulnérables d'entre nous.

Les premières conséquences du confinement observées sur le terrain, dans mon département comme ailleurs, sont sans appel : anorexie et amaigrissement, déclin cognitif accéléré, majoration de troubles du comportement, tristesse, etc. Parmi les recommandations de nos rapporteurs, nous retiendrons le renforcement des outils de gestion des risques en établissements médico-sociaux, l'élargissement du plan Bleu, conçu à l'époque pour le risque canicule, la systématisation de l'élaboration des plans de continuité de l'activité (PCA) ou encore l'intégration automatique des Ehpad et des autres établissements sociaux et médico-sociaux aux exercices annuels organisés sur la gestion des risques. Enfin, il conviendrait d'accroître la couverture des Ehpad par des médecins coordonnateurs, de donner à ces derniers un rôle plus affirmé de chef d'orchestre

Chevrollier. Je remercie d'abord l'ensemble des collègues qui ont participé à la mission de contrôle dans le cadre de cette commission d'enquête sur la gestion de la crise covid-19, qui dure malheureusement toujours. Ils ont accompli un travail minutieux et complet qui a permis de mettre en lumière les causes de l'impréparation de nos politiques publiques face à la crise sanitaire de révéler un certain nombre de difficultés, voire de dysfonctionnements de notre système de santé. Monsieur le ministre, j'évoquerai le problème récurrent de la démographie médicale. Au pic de la crise du covid-19, des infirmières issues d'autres spécialités ont dû se former en urgence aux gestes de réanimation. Des internes de première année ont assumé des responsabilités de niveau troisième ou quatrième année. J'ajoute que l'on manque de médecins et de spécialistes et que des départs à la retraite ne sont pas compensés. constate un vieillissement de la population, des exigences de plus en plus fortes des patients et les besoins de santé sont appelés à augmenter. Le problème de la démographie médicale touche tous les territoires, notamment les plus ruraux, et concernerait une commune sur trois. Tous les trois ans est présenté un projet de loi santé ou un plan gouvernemental traitant en partie de cette question. Pourtant, le nombre de Français privés de médecin traitant atteindrait près de 7,5 millions de personnes, soit 11 % de la population. C'est un véritable sujet d'inquiétude pour nos concitoyens et pour les élus. La campagne de vaccination débute, mais elle n'est pas accessible aux patients qui n'ont pas bénéficié d'une consultation médicale. Comment feront tous ceux qui n'ont pas de médecin traitant ? Comment mener une campagne efficace dans ces territoires qui sont loin des hôpitaux et des centres de vaccination ? Le rapport de la commission d'enquête fait état d'une logique française hospitalo-centrée : « Si les lacunes de la liaison ville-hôpital se sont faites cruellement sentir, des initiatives de coopération entre acteurs, souvent isolées, sont des atouts sur lesquels capitaliser. L'organisation des soins doit donc s'établir en collaboration avec les élus locaux et la médecine de ville pour répondre aux besoins des territoires et à la demande des patients dans le cadre d'un parcours de soins. Monsieur le ministre, quelles solutions proposez-vous pour assurer une meilleure répartition

L'heure n'est pas encore au bilan », a indiqué le ministre de la santé en réponse aux premiers orateurs de notre débat. C'est sans doute pourquoi sa réponse a été si brève, témoignant à l'évidence d'une certaine lassitude à devoir rendre compte devant le Parlement, malgré l'amour proclamé à son endroit. Monsieur le ministre, vous avez cité Churchill. Permettez-moi de vous citer Shakespeare : « Il n'y a pas d'amour ; il n'y a que des preuves d'amour. » Répondre aux parlementaires peut en être une.

Je regrette notamment que vous n'ayez pas répondu sur la question de l'isolement, question qui me semble encore ouverte, et, plus généralement, sur la stratégie « tester, tracer, isoler » et les raisons pour lesquelles elle est devenue « tester, alerter, protéger

les Allemands ont su financer des biotechs, mais la France ne parvient pas à financer les siennes et, surtout, à fidéliser ses chercheurs. La temporalité a été évoquée, monsieur le ministre, ainsi que le temps long. J'entends ces arguments, mais, au printemps les Français n'ont pas compris pourquoi, en dépit des déclarations du Gouvernement, ils n'avaient pas de masques. Il était de notre devoir- et je ne dis pas seulement du vôtre -de chercher à comprendre, d'autant que, dans ce domaine, la stratégie et le discours ont clairement été dictés par les capacités. Sur ce dossier, le de la commission d'enquête, à l'issue de la première vague, était le bon : nous ne parlons plus de masques aujourd'hui. Non, monsieur le ministre, sur les masques, la commission d'enquête ne s'est pas focalisée sur un nombre ; elle a proposé une méthode et un schéma d'organisation, ce qui est très différent. Je récuse l'accusation de politique politicienne. Vous n'en trouverez pas trace dans le rapport. Par ailleurs, j'entends bien que les tests sont gratuits, mais cela ne rend pas pour autant leur usage efficace pour casser les chaînes de contamination. Nous ne tirerons les leçons de la crise qu'à condition d'accepter d'entrer dans la logique du débat. À l'évidence, ce travail reste à faire. Fort heureusement, et je vais rebondir sur une réponse que vous avez donnée sur un ton un peu énervé ... Je ne me suis pas énervé ! Fort heureusement, monsieur le ministre, le contrôle de l'action du Gouvernement et de l'administration ne se fait pas uniquement devant les tribunaux. La commission d'enquête n'a jamais- jamais -appelé à traduire quiconque devant une cour de justice. Elle a seulement appelé à changer un mode de fonctionnement : une véritable agence sanitaire ne voit pas ses conclusions modifiées par le directeur d'une administration centrale. est le sens de nos recommandations et je n'accepterai pas, sur ce sujet en particulier, de caricature. Nous en avons

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que l'épidémie de covid-19 sévit depuis bientôt un an en France, une partie des victimes indirectes reste largement oubliée : les étudiants. Devant la situation très préoccupante qu'ils vivent quotidiennement et l'absence de réaction suffisante du Gouvernement, nous avons souhaité mettre ce sujet à l'ordre du jour. Nous voulons alerter et proposer des mesures rapides et concrètes, face à la montée de la précarité et des risques psychosociaux qui épuisent notre jeunesse. Cela fait plusieurs semaines que les témoignages affluent. Les étudiants et les étudiantes veulent se faire entendre et nous disent combien leur situation s'est dégradée matériellement et, plus inquiétant encore, mentalement. La crise sanitaire a fait ressortir l'état de délabrement déjà existant des universités. La question est posée : que pouvons-nous proposer à nos jeunes pour améliorer leurs conditions de vie et d'études, particulièrement dans le contexte sanitaire actuel, mais aussi à plus long terme ? Quelles perspectives voulons-nous offrir à notre jeunesse ? Les chiffres publiés ces derniers mois sont effrayants : selon un sondage de la Fondation Abbé-Pierre, 20 % des jeunes ont eu recours à l'aide alimentaire au cours de la crise sanitaire.

seulement 36,8 % des étudiants ont touché des bourses sur l'année scolaire 2019-2020, celles-ci ne permettent souvent pas de vivre sans travailler à côté. Or le cumul entre études et emploi est la première cause d'échec à l'université. À cette précarité grandissante s'ajoute le poids de l'isolement devant les écrans. Il en résulte un enseignement désincarné, sans contact humain, face auquel les étudiants peinent à suivre le rythme et à conserver leur motivation. Pour beaucoup, c'est la même journée qui se répète, comme en témoigne Marva, étudiante à Toulouse : « Réveil à 7 heures 30, 8 heures d'écran par jour, repas, révisions, dodo. Au début, on se dit que ça va aller, et puis on finit par craquer. Selon une étude réalisée auprès de 70 000 étudiants lors du premier confinement, 43 % des étudiants sont affectés par un trouble de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression. Face à cela, les services de santé universitaire sont totalement saturés. Tout cela engendre un manque de perspective pour les étudiants. Les risques de décrochage ou de non-validation de l'année universitaire les inquiètent, mais aussi les stages annulés, l'entrée sur un marché du travail tendu ou encore l'impossibilité de partir étudier à l'étranger. À un âge où, d'habitude, l'on prend son envol, de nombreux étudiants sont rentrés chez leurs parents. Pour les enseignants, cette situation est également très difficile. Comment donner des cours interactifs face à une mosaïque d'écrans noirs ? Comment intéresser des étudiants qu'ils n'ont parfois jamais rencontrés et dont ils devinent les difficultés sans avoir pour autant les moyens de les identifier et de les aider ? Le personnel administratif est lui aussi obligé de faire et défaire depuis des mois, pour organiser les emplois du temps, en distanciel, puis en présentiel, tout en respectant des directives changeantes et imprécises, qui ne sont pas forcément adaptées aux réalités du terrain. Il faut avouer que le décalage entre les protocoles sanitaires nous interpelle. Les commerces et les écoles sont restés ouverts ; les étudiants en classes préparatoires et en BTS suivent des cours normalement. Il y a une différence de traitement évidente et les étudiants à l'université se sentent, à juste titre, laissés pour compte.

Seuls 10 restaurants universitaires étaient ouverts sur 27 et il était impossible de prendre les repas sur place. Sous la pluie, les étudiants se regroupaient dans des voitures, alors que la surface du restaurant universitaire aurait permis de mieux respecter les gestes barrières. Là aussi, les ordonnances venues d'en haut étaient aveugles à la réalité du terrain, créant des risques sanitaires supplémentaires qui doivent être évités. Depuis votre annonce, vendredi dernier, permettant la restauration sur place, je suis soulagée, mais, encore une fois, cela aurait pu être envisagé plus tôt D'autres mesures sont positives, bien sûr, telles que la création de étudiants, le recrutement d'assistantes sociales et de professionnels de santé universitaire ou encore le chèque de santé mentale, même si la démarche pour en bénéficier est compliquée.

Selon la totalité des collectifs et syndicats étudiants que nous avons rencontrés, ces mesures sont loin d'être suffisantes. En effet, la covid-19 a aggravé une situation qui était déjà critique en matière de pauvreté des étudiants, d'échec à l'université et de manque de moyens généralisé. À quand une réponse structurelle à ce problème, pour donner à tous les étudiants les meilleures conditions pour réussir leurs études ? Dans les pays scandinaves, chaque étudiant perçoit une allocation individuelle, indépendamment du revenu de ses parents, pour lui permettre de se consacrer sereinement à ses études et de prendre son autonomie.

cette plaie qui mine notre société française au système scolaire inégalitaire. Avec l'allocation d'autonomie, on reconnaît les étudiants comme des adultes à part entière. C'est aussi un autre rapport qui se noue entre l'État et ces jeunes, un rapport fondé sur la confiance. Madame la ministre, nous vous demandons solennellement d'entamer une véritable réflexion sur ce sujet. Désireux de s'inscrire dans une démarche constructive et durable, les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ont écrit un courrier au Premier ministre, qui vous a été également transmis. Dans ce Dans ce courrier, nous appelons à un plan massif d'investissement dans les universités, pour soutenir la jeunesse sur le court et le long terme, autour des grands axes suivants. Cela passe par l'égalité de traitement entre tous les étudiants, qu'ils soient en classes préparatoires aux grandes écoles, en BTS ou à l'université, le retour en cours à 50 % des étudiants, avec des moyens humains et techniques pour permettre un dédoublement des groupes et des cours hybrides- cours présentiels diffusés aussi à distance -, en faisant confiance à la communauté universitaire pour s'organiser au mieux, en fonction des contraintes et des possibilités du contexte. une sécurité financière accrue, avec une aide d'urgence pour tous les étudiants, ainsi qu'une revalorisation significative des bourses et de l'aide personnalisée au logement (APL), comme par des investissements sanitaires massifs dans les locaux universitaires, en matière de ventilation et d'équipement numérique. l'inclusion de tous les étudiants, avec une adaptation des examens à la situation sanitaire et l'assurance qu'aucun étudiant ne sera pénalisé en raison de l'épidémie. une politique de recrutement sanitaire ambitieuse, pour garantir un nombre suffisant d'assistantes sociales et de professionnels de santé auprès des étudiants- pour le moment, le compte n'y est pas

Madame la ministre, nous connaissons les efforts financiers importants que le Gouvernement a consentis depuis le début de la crise. Aujourd'hui, nous vous demandons de continuer ces efforts envers notre jeunesse et d'entendre réellement ses cris d'alarme.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis le début de la crise sanitaire, dans cet hémicycle, nous alertons le Gouvernement sur les conditions de vie et d'études de nos étudiants. Je remercie nos collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires d'avoir demandé l'inscription de ce débat à l'ordre du jour À chaque prise de parole, les mêmes mots reviennent comme une insupportable antienne : angoisse, désespoir, solitude, isolement, précarité. L'Observatoire national de la vie étudiante décrivait, dès avant le second confinement, une nouvelle dégradation des conditions d'études et de santé 31 % des étudiants présentaient déjà des signes de détresse psychologique. Signe que ce sujet demeure prégnant, les commissions d'enquête, les missions d'information et les débats se multiplient à l'Assemblée nationale comme au Sénat afin de trouver des solutions à la crise que les étudiants une crise dont les emmurés de vingt ans subissent pleinement les effets sans en être pour autant les victimes directes. Bien évidemment, on peut saluer les annonces du Président de la République, l'accès aux repas à 1 euro du Crous et à une consultation gratuite auprès d'un psychologue ou encore la reprise partielle des enseignements en présentiel. Ces mesures donnent une bouffée d'oxygène, elles évitent la catastrophe. Madame la ministre, est-ce pour autant suffisant ? Je ne le crois pas. Nos étudiants ne veulent pas que l'on s'apitoie sur leur sort. Ils veulent savoir où on les conduit. Je crois en effet que l'une des principales causes de ce mal-être est bien l'angoisse générée par un pilotage à vue,

Le 14 janvier dernier, c'est une reprise des enseignements à 50 % qui se dessinait, uniquement pour les travaux dirigés et les apprentis. Aujourd'hui, la jauge est fixée à 20 % maximum. Comment voulez-vous que l'on s'y retrouve ? Les étudiants, les enseignants et le personnel universitaire sont usés par cette incapacité à tracer des perspectives et à s'y tenir. Lassés, ils demandent désormais le maintien des conditions actuelles d'enseignement

Cette angoisse se nourrit également d'incompréhensions et de découragement. Comment comprendre la différence qui est faite entre les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections de technicien supérieur d'un lycée, Au-delà, comment les uns et les autres peuvent-ils comprendre qu'ils paient un si lourd tribut à la gestion d'une épidémie qui ne les affecte qu'à la marge ? Comment peuvent-ils envisager leur avenir, quand leur vie et les outils nécessaires à leur construction sont mis sous cloche ? Aujourd'hui, ils se sentent non essentiels, lâchés et abandonnés par la génération du « Il est interdit d'interdire », celle-là même qui leur interdit de sortir après dix-huit heures. Je ne nie pas la nécessité de respecter sur les campus comme ailleurs les indispensables gestes barrières. Je dis simplement qu'un peuple majeur et sa jeunesse ont besoin d'explications et de cap. Je dis simplement que les universités et les établissements d'enseignement supérieur ont besoin de la confiance du Gouvernement. Je dis qu'ici comme ailleurs nous sommes victimes d'une gestion par trop centralisée. Il est donc impératif de laisser de la marge aux universités, pour qu'elles s'organisent dans l'objectif d'accueillir autant d'étudiants que possible. Il est impératif de leur permettre d'évaluer, site par site, leur capacité d'accueil afin d'établir des jauges adaptées. jauge de 20 % n'est-elle pas en effet contreproductive, quand les salles ou les sites sont suffisamment grands pour accueillir plus de 20 % d'étudiants Permet-elle suffisamment d'optimiser le nombre de personnes dans les 18,5 millions de mètres carrés des locaux universitaires ? Ici comme ailleurs, madame la ministre, il est temps de faire confiance aux universités et de vous appuyer sur leur agilité et leur proximité pour redonner espoir et confiance en leur avenir aux jeunes de ce pays. Voilà, madame la ministre, les interrogations que je vous livre. Au-delà des mesures d'accompagnement annoncées par le Président de la République, envisagez-vous de faire confiance au terrain et de lui donner de la liberté, pour qu'il puisse s'adapter aux réalités ? Faites confiance aux responsables des universités et des établissements d'enseignement supérieur ! Ils sont, sur le terrain, mieux armés pour lutter contre ce terrible mal-être qui ébranle la jeunesse de notre pays ! La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant la crise sanitaire, la précarité étudiante était déjà une réalité. Près d'un étudiant sur deux travaillait pour financer ses études et subvenir à ses besoins. L'accès au logement, aux soins et à une alimentation saine constituait un défi quotidien pour bon nombre de nos étudiants. L'action gouvernementale reposait alors sur trois leviers complémentaires : l'augmentation des bourses sur critères sociaux, la construction de nouveaux logements universitaires et la mobilisation d'aides pour les situations d'urgence. Depuis le 14 mars 2020, la décision du Gouvernement de fermer les établissements d'enseignement supérieur pour protéger la population du covid-19 a changé la donne. Depuis lors, les situations de précarité que nous connaissions avant la crise s'aggravent et se multiplient. La moitié des étudiants qui travaillaient pour vivre ont perdu leur emploi. À cela s'ajoute la détresse psychologique liée à l'isolement social d'une grande partie de notre jeunesse. L'étude menée à ce sujet par l'Observatoire national de la vie étudiante en dit long : 31 % des étudiants interrogés ont connu une détresse psychologique lors du confinement. S'y ajoutent aussi les incertitudes qui pèsent sur l'avenir des futurs diplômés. L'accès aux stages, dans un tel contexte de crise sanitaire et économique, est fortement menacé. La constitution des futurs réseaux professionnels l'est tout autant. Nous connaissons des risques accrus de décrochage scolaire, notamment en première année de licence. Tout n'est pas perdu : l'apprentissage a connu un engouement inédit l'année dernière, malgré la crise, avec la signature de 500 000 contrats. Le plan de soutien à l'apprentissage du Gouvernement y est pour beaucoup. Notre groupe est très favorable à la prolongation de ce dispositif qu'a annoncée la ministre du travail, Mme Élisabeth Borne. Les mesures palliatives prises par le Gouvernement constituent des gestes plus ou moins importants : les repas à 1 euro pour tous, l'accès au soutien psychologique et, surtout, le retour progressif aux cours en présentiel, puisque c'est bien le véritable sujet, madame la ministre. Les étudiants demandent à étudier dans de bonnes conditions, à retrouver le lien avec leur université, leurs professeurs, leurs camarades. L'émulation qui se rencontre au sein des campus est irremplaçable. je partage l'avis du professeur Delfraissy : le retour en cours des étudiants est une question de santé publique. Nous devons aussi veiller à la bonne lisibilité de l'action publique et, pour cela, assurer une cohérence entre les différentes décisions. cette question : comment justifier la fermeture des universités, par prudence, alors que les classes préparatoires et les classes de BTS restent ouvertes ? Les étudiants demandent que leur avenir ne soit pas sacrifié ; ils demandent surtout à être écoutés et pris en considération. dernier, le Président de la République a annoncé une reprise partielle des cours en présentiel. Nous devons favoriser la souplesse des dispositifs. De nombreux étudiants ne pourront pas revenir étudier en présentiel un jour par semaine, faute de logement. faisons confiance aux jeunes qui sont l'avenir de notre pays ! Ne les infantilisons pas, ne condamnons pas leur avenir ! Des milliers de jeunes enfants sont actuellement regroupés en classe maternelle ou en école élémentaire ; ils partagent la même table de restauration collective, Les jeunes adultes qui peuplent nos campus universitaires et nos grandes écoles sont, à mon sens, capables d'être responsables et de respecter les gestes barrières. Si le risque n'est pas dans les amphithéâtres, où les étudiants seront masqués et distanciés, pourquoi ne pas limiter l'accès des restaurants universitaires aux repas à emporter ? Ce sont des centaines de milliers de jeunes qui baissent les bras et risquent d'abandonner leurs études. Nous devons trouver des solutions à court terme et à long terme pour faciliter la résilience de la jeunesse et éviter qu'elle ne paie, sous une autre forme, un lourd tribut à l'épidémie. N'oublions pas qu'elle est la richesse de la France de demain ! La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Monique de Marco vous a présenté, dans sa globalité, l'analyse et le regard des écologistes sur la crise majeure qui bouleverse le monde étudiant de notre pays. ma part, je m'attarderai sur un point particulier qui me semble essentiel : la santé mentale des étudiants. La détresse psychologique des étudiants a été une dimension sous-estimée de la crise que traverse la jeunesse. De récentes tentatives de suicide ont jeté une lumière crue sur la détresse qui frappe de nombreux étudiants et étudiantes. On le sait, la série de restrictions que nous impose la crise sanitaire frappe durement la jeunesse : absence de vie sociale, arrêt des cours en présentiel, cantonnement des étudiants dans leurs logements parfois vétustes, impossibilité de mener d'autres activités ou de travailler, autant de difficultés qui viennent sérieusement amplifier les problématiques de santé mentale.

En réalité, la jeunesse compte plus d'un million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. En réalité, une génération entière voit ses perspectives disparaître à l'ombre des crises économiques, sociales et, bien sûr, climatiques.

Il y a un an, il était tout à fait nécessaire de prendre des règles de confinement d'urgence. Tous les campus ont été fermés, comme le reste du pays. Un an plus tard, il est temps de travailler à des protocoles sanitaires de crise adaptés, des protocoles pensés en fonction des campus, des universités et de leurs capacités, et non plus fixés uniformément pour toute la France, à des protocoles qui doivent permettre le retour d'étudiantes et étudiants en présentiel, même partiellement. Trouvons enfin des solutions, maintenant, pour celles et ceux qui sont en détresse psychique, pour celles et ceux qui ne peuvent plus continuer leur vie comme avant Les conséquences du 100 % distanciel sur l'état psychologique des étudiants ont été largement sous-estimées. Il faut de l'accompagnement humain. Or, dans ce domaine, la France est en queue de classement par rapport aux autres pays développés, et de très loin

La Charte de l'accréditation internationale des services de santé mentale universitaire recommande de viser un taux de 1 psychologue pour 1 000 à 1 500 étudiants. Si aucun pays n'atteint à ce jour ce chiffre ambitieux, force est de constater que la France en est loin, très loin. En janvier dernier, le Gouvernement a annoncé vouloir doubler ce chiffre, en recrutant 80 psychologues universitaires, portant ainsi le ratio à 1 psychologue pour 15 000 étudiants. Cet effort doit être salué, bien sûr, mais comme de nombreuses réformes entreprises par ce gouvernement en direction de la jeunesse, nous avons un souci d'échelle. Ainsi, la création d'un « chèque psy » s'inscrit dans cette même démarche. Ce chèque, qui porte mal son nom puisqu'il s'agit en réalité de séances gratuites, permettra aux étudiants de bénéficier de trois rendez-vous chez un Mais comment satisfaire cet objectif louable alors que notre pays est si dramatiquement sous-doté en termes de personnel qualifié ? Afin de commencer à avoir un accompagnement correct dans tous les services universitaires, encore nous faudrait-il atteindre le ratio de 1 psychologue pour 4 000 étudiants, ce qui implique le recrutement de 520 psychologues. Nous en sommes loin Il s'agit non pas d'appeler à une dépense inconsidérée ni de céder à un caprice électoraliste, mais, au contraire, de répondre à l'urgence réelle et terrifiante des files d'attente qui s'allongent devant les bureaux des psychologues universitaires, et à celle des 22 % d'étudiants qui ont eu des pensées suicidaires. Il s'agit d'investir d'urgence dans l'avenir de notre jeunesse

Investissez dans les campus afin de permettre le retour des étudiants en présentiel, investissez dans les aides matérielles et financières indispensables à la poursuite des études, investissez dans la création de postes de psychologues ! Regardez enfin la jeunesse en face, permettez-lui d'envisager son avenir avec espoir ! La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le lundi 1 février 2021, nous vous recevions, madame la ministre, sur le domaine universitaire de Bordeaux, pour vivre ensemble la rentrée d'une poignée d'étudiants qui faisaient leur retour sur un campus bien désert. Ces initiatives sont encourageantes ; elles sont importantes pour le moral de certains jeunes, mais tous ne peuvent y accéder. En effet, beaucoup de jeunes, malgré l'aide de leur famille, n'ont pas eu les moyens de continuer à louer un appartement et assumer le coût de la vie dans nos grandes villes, ce dès le mois de décembre. Un retour obligatoire en présentiel doit être organisé à l'avance, pour ne pas créer de nouvelles difficultés. L'année universitaire étant désormais sérieusement avancée, il serait raisonnable de donner des perspectives claires à nos étudiants. Il conviendrait surtout que vous leur annonciez que c'est avec eux que vous allez construire les conditions de leur retour. Avec eux, parce que nos jeunes font preuve de responsabilité ; ils n'ont jamais été aussi conscients de la gravité de la situation, aussi respectueux des règles établies, aussi volontaires dans l'effort. Mais ils n'ont jamais été aussi mal

nous ne pourrons pas le justifier, nous le pourrons plus ! Très bien ! C'est le prix de notre responsabilité vis-à-vis d'une classe d'âge qui se morfond. Madame la ministre, vous disiez à ces jeunes qu'ils pourraient raconter, dans quelques années, qu'ils ont participé à un effort nécessaire pour le pays, et vous aviez raison. Nous leur en sommes bien sûr reconnaissants, mais au prix de quels renoncements ? Celui de voir notre jeunesse inemployée, paupérisée, isolée et dépressive ! Nous sommes à la limite de créer les conditions d'un affaiblissement durable de notre nation, en effritant la résilience de ce qui fait son corps social, l'énergie jusqu'alors inébranlable des hommes et des femmes qui nous entourent, leur capacité à affronter le réel, à surmonter les crises, à prendre conscience que les pandémies et les guerres existent, et que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Nos jeunes ne disposeront pas de ces clefs si nous les laissons durablement dans l'éther d'un monde figé face au risque. La plus grande preuve d'amour que nous puissions leur donner est de leur permettre de « revenir du familier à l'étrange et, dans l'étrange, affronter le réel », comme l'écrivait Paul Valéry. Car, en attendant, leur réel est moins l'exposition au virus que l'isolement, la désolation et la rupture. L'accompagnement psychologique que nous avons vu s'exercer à Bordeaux, lors de votre venue, est indispensable. Le modèle des « sentinelles », ces jeunes qui sont formés pour accompagner les autres en détectant les signes pathologiques faibles, est un bon modèle, quoique insuffisant à ce stade.

Toutes celles et tous ceux qui avaient un job étudiant en plus de leurs études se trouvent pénalisés par la fermeture de nombreux établissements et l'annulation d'événements. Aussi, je tiens à saluer les initiatives locales prises par les municipalités, les universités, les Crous et les banques alimentaires, ainsi que par tant de bénévoles des associations

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, samedi dernier, à Bagneux, je participais à une collecte alimentaire au profit des étudiants de cette commune populaire de mon département. Des personnes aux revenus très modestes donnaient ce qu'elles pouvaient, émues par les images de ces longues files d'étudiants attendant une pitance devenue leur seul repas quotidien. La solidarité est souvent exercée par les pauvres pour les plus pauvres qu'eux. Je garde en mémoire l'image de cette femme au panier de courses à peine rempli, offrant un paquet de pâtes, en me demandant comment il était possible que, dans notre pays, une personne accédant à l'université puisse souffrir de la faim. de la faim. En 2019, par la loi de finances rectificative, votre gouvernement avait supprimé 35 millions d'euros de crédits du programme « Vie étudiante ». En 2018 et 2019, ce sont 100 millions d'euros de crédits votés par le Parlement

des moyens d'urgence leur permettant d'aider rapidement les étudiants. Par la voix de M. Darmanin, alors ministre de l'action et des comptes publics, le Gouvernement m'avait expliqué que des crédits budgétaires supplémentaires La politique du « quoi qu'il en coûte » a ignoré les campus et la détresse estudiantine. Cet automne, nous avons discuté d'une loi de programmation de la recherche, qui nous a été présentée par le Gouvernement comme le plus gros effort budgétaire depuis la Libération. L'université n'a bénéficié dans ce cadre d'aucune aide budgétaire supplémentaire, comme si les étudiants d'aujourd'hui n'étaient pas les chercheurs de demain ... J'entends en ce moment les déclarations compassionnelles du Gouvernement, qui s'alarme du mal-vivre des étudiants. La pandémie n'en est pas l'unique cause : dans les universités, comme à l'hôpital, la crise sanitaire est révélatrice d'une situation de sous-investissement chronique, qui a fragilisé tout le service public de l'enseignement supérieur. Certes, l'état de carence de l'université n'est pas imputable à votre seul gouvernement. Cela fait une vingtaine d'années que l'État n'investit plus dans l'enseignement supérieur, et que l'université est soumise aux ciseaux malthusiens d'une hausse continue du nombre d'étudiants et d'une stagnation de ses budgets. Le budget moyen alloué à chaque étudiant ne cesse de baisser depuis dix ans ; cette année, il devrait même passer sous le seuil symbolique des 10 000 euros. En revanche, le budget moyen consacré aux étudiants des classes préparatoires n'a cessé d'augmenter, atteignant bientôt 16 000 euros. Voilà Voilà votre choix politique ! Cela fera bientôt quatre ans que votre gouvernement gère, avec tous les pouvoirs, les affaires de notre pays : l'heure des bilans Dans le domaine de l'enseignement supérieur, la politique menée par votre ministère ne se distingue en rien de celle menée par tous ceux qui vous ont précédée. Elle n'a fait qu'accompagner un progressif, mais irrépressible, désengagement de l'État. L'université n'a pas été une priorité politique de votre gouvernement ! Les premières victimes de ce sous-investissement chronique sont les étudiants. Avant la crise, leur situation matérielle ne leur permettait pas de poursuivre leur cursus dans de bonnes conditions pédagogiques ; avec la crise, ils souffrent d'une paupérisation dramatique, qui s'ajoute à l'isolement, la privation de vie sociale, à l'absence de toute perspective, avec une inquiétude grandissante sur la valeur qui sera attribuée à leur diplôme. Avant la crise, 40 % des étudiants travaillaient pour financer leurs études avec la crise, près de 60 % d'entre eux ont été privés de toute activité salariale. Le Président de la République a affirmé qu'un étudiant devait avoir les mêmes droits qu'un salarié. Pourquoi ne profitent-ils donc pas des mesures de chômage partiel pour toutes ces activités salariées qui les faisaient vivre et qu'ils ne peuvent plus exercer ? Les étudiants n'en peuvent plus de souffrir de la faim, de la réclusion, du sentiment d'abandon, de la privation de tout ce qui faisait le bonheur d'être jeune, et plus encore

étudiant disait : « La vraie honte, c'est de voir tant d'étudiants peinant à se nourrir, alors qu'en se formant, ils créent la richesse de demain. » La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « on veut un amphi, pas un psy ! » : tel est le cri des étudiants français en ce début d'année 2021, après un an de fonctionnement des universités sur un mode très dégradé. C'est en échangeant avec des étudiants, en écoutant leurs témoignages, que cette phrase a retenu toute mon attention, et a pris tout son sens. Il y a un mois environ, lors de la séance de questions d'actualité au Gouvernement, je vous interrogeais, madame la ministre, sur la détresse des étudiants,

Le désenchantement est d'autant plus grand que les étudiants en master vont entrer sur un marché du travail en crise, où la perspective d'une évolution sociale permise par l'accomplissement d'études supérieures s'amenuise.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, de juin dernier, la sociologue Anne Lambert alertait sur la gravité spécifique de la crise pour les jeunes. À la fois révélatrice des maux et des inégalités qui les frappent depuis de nombreuses années, elle a pour effet de les décupler, au point de dégrader plus encore les conditions d'insertion dans la vie adulte. Sa préconisation se révélait donc sans appel : « On a longtemps pensé que l'âge de la jeunesse pourrait ouvrir l'éventail de la reproduction sociale et élargir l'espace des possibles : cette illusion tombe, les cartes ne sont pas rebattues. Pour aide les jeunes, et notamment les plus précaires, il faut une réponse massive et d'envergure de la part des pouvoirs publics.

Quant aux constats, si nous pressentions- bien plus que nous ne mesurions ! -l'impact désastreux de la crise sur les jeunes à l'époque, les effets sont désormais visibles, quantifiables et analysables, de telle sorte qu'il est impossible d'ignorer l'urgence d'agir.

Ainsi, aux trois cassures, pédagogique, économico-sociale et psychologique, du premier confinement répondent aujourd'hui trois risques de rupture identiques. En premier lieu, la rupture académique peut encore être évitée en s'assurant que l'année universitaire 2020-2021 ne soit pas une année blanche. Il s'agit d'appliquer le mantra selon lequel « il faut sauver le second semestre », et permettre à tous les étudiants d'être, au maximum, et en fonction de la circulation du virus, en présentiel. La jauge actuellement fixée à 20 %, soit un jour de présence par semaine, constitue un premier pas, mais il est primordial qu'il ne soit pas le dernier.

Les établissements pourront ainsi être plus réactifs et adapter les protocoles aux situations spécifiques de chaque campus. Madame la ministre, faites-leur confiance

Sans prétendre à l'exhaustivité, trois problématiques se posent avec acuité pour le second semestre. Tout d'abord, il est nécessaire de disposer d'un cadre pour les évaluations, par-delà les incitations et les incantations. Les étudiants ont en effet besoin d'un cadre stabilisé, protecteur et rassurant, qui tienne compte du contexte actuel, et ne soit pas générateur de stress ni d'angoisse. Il nous faut aussi réfléchir à un mécanisme compensatoire pour les étudiants qui n'auront pas pu réaliser leur stage. Enfin, il est indispensable de soutenir les enseignants et enseignants-chercheurs qui, pour beaucoup, ont mis entre parenthèses leurs travaux de recherche.

inacceptable, à l'image de la précarité menstruelle, qui toucherait une étudiante sur trois ! Au fond, l'évolution est en miroir de celle que traverse la société dans son ensemble. Des étudiants qui n'étaient pas dans une situation financière délicate avant la crise sont en train d'y tomber. Deux publics en particulier semblent très vulnérables : les étudiants internationaux-

Néanmoins, des acteurs de terrain et des étudiants nous font part de l'existence de deux écueils principaux. Le premier a trait à l'absence de stratégie globale pour lutter contre la précarité étudiante. Si les aides ponctuelles sont bienvenues- je m'en félicite -, elles ne constituent pas pour autant une réponse durable et synoptique au défi actuel. Leur caractère ponctuel et éclaté apparaît en décalage avec le nécessaire accompagnement financier sur le temps long, dont bon nombre d'étudiants ont besoin, y compris ceux étant à la recherche d'un premier emploi. À cet égard, il est assez étonnant que vous ayez supprimé l'aide à la recherche du premier emploi,

Comme pour les autres domaines, il est urgent de simplifier les procédures, et de renforcer les équipes, notamment au sein des Crous et des services universitaires de santé. Nous ne pouvons ni accepter ni nous résoudre à cette paupérisation croissante des étudiants, nous ne voulons pas que la jeunesse soit exsangue au sortir de la crise ! Nous devons agir sur deux échelles.

et incompréhensible, dans une période aussi tragique pour les jeunes, qu'une réforme plonge certains d'entre eux plus encore dans la précarité et le désarroi à plus long terme et de façon plus structurante, nous réitérons notre demande d'ouvrir le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) dès 18 ans, conformément à la proposition de loi déposée par notre groupe, et de mener une consultation approfondie pour la mise en oeuvre d'une allocation d'autonomie pour chaque jeune. Que cette crise nous permette au moins de repenser l'émancipation et l'insertion dans la vie active de notre jeunesse ! La rupture psychologique, quant à elle, dérive des deux précédentes ; elle en est même la conséquence directe. Passez-moi l'expression, mais les chiffres font froid dans le dos ! Près de 800 000 étudiants présenteraient un état de souffrance psychique ; 11,4 % des 70 000 étudiants interrogés par le Centre national de ressources et de résilience (CN2R) ont cultivé des idées suicidaires- et que dire des drames survenus ces derniers mois L'isolement pesant depuis près d'un an et l'amoncellement des difficultés, qu'elles soient financières, sociales, académiques ou administratives, finissent vraiment par fragiliser dangereusement la santé mentale des étudiants. Il faut aussi le préciser, l'épidémie actuelle révèle au grand jour les failles de notre système de soins, qui a toujours été plus tourné vers le curatif que le préventif. Or les manques de notre politique de prévention se font aujourd'hui ressentir.

est une bonne mesure. Il faut que le dispositif soit simple d'accès pour l'étudiant. Beaucoup de professionnels nous ont alertés sur l'absolue nécessité de ne pas limiter ce chèque à trois consultations, le suivi psychologique d'un étudiant requérant parfois plus de rendez-vous.

cette jeunesse qui a accepté de mettre sa vie entre parenthèses pour protéger les plus vulnérables, nous sommes profondément redevables. Et nos obligations, notre devoir collectif à son égard iront au-delà de la crise sanitaire. La réparation que nous lui devons s'inscrira dans une durée bien plus longue ; elle devra être à la hauteur de l'abnégation de ces jeunes. Notre exigence, que j'espère commune, sera de nous souvenir, de permettre une réparation juste, de composer de nouveaux espoirs. Car l'esprit de responsabilité dont ces jeunes font preuve aujourd'hui

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, concertation, stabilité et cohérence : voilà ce que souhaitent les étudiants et la communauté enseignante ; voilà ce dont a besoin l'université Les efforts consentis par nos étudiants en cette période de crise sanitaire sont immenses. Ne connaissant finalement que peu de formes graves de la covid-19, ils sont soumis à des restrictions rigoureuses de leur mode de vie, entraînant pour beaucoup une grande précarité. D'innombrables témoignages illustrent cette détresse étudiante. À cela s'ajoute l'incertitude face à l'avenir. Notre jeunesse, considérée comme inébranlable, montre aujourd'hui les stigmates d'un combat qu'elle ne peut pas supporter à elle seule. Les récentes annonces du Président de la République, même si elles prennent en compte une partie des revendications, ne peuvent pas être considérées comme suffisantes. Ces mesures d'accompagnement ont été mises en oeuvre en réaction à la crise étudiante. Et c'est ce manque d'anticipation qui plonge dans le désarroi des milliers de jeunes. Rappelons l'action dynamique et concrète des collectivités. Je le constate notamment dans mon territoire. Région Sud, le département des Alpes-Maritimes et les communes sont mobilisés de toutes leurs forces pour le bien-être des étudiants. La métropole Nice Côte d'Azur présente en ce moment même de nouvelles actions. Le village de Gilette, quant à lui, organise une collecte pour leur venir en aide. Sur le terrain, je dialogue régulièrement avec des étudiants et des membres de la communauté enseignante. Ces échanges m'ont amenée à alerter rapidement le Gouvernement, puis à proposer la demande de reprise, à hauteur de 50 %, ainsi que l'accélération et la systématisation de l'offre de vaccination pour les volontaires. L'université passe avant tout par des interactions entre professeurs et étudiants. Couper ce lien, c'est donc amoindrir l'envie que les étudiants ont de se lever tous les jours pour apprendre. Rétablir un rythme de travail à 50 %, que les cours à distance ont tendance à diluer, permettra de sortir les étudiants de l'isolement et d'une solitude où s'érode jour après jour leur motivation. Limiter à 20 % le présentiel ne permet pas de résoudre toutes les inégalités. Il faut poursuivre les efforts. technicien supérieur (BTS) et à l'université ont les mêmes droits, mais ne bénéficient pas des mêmes conditions garanties par l'État. Et c'est notamment cette différence de traitement qui suscite l'incompréhension. En quoi ce brassage serait-il différent ? Je crois qu'il faut cesser cette infantilisation, qui sacrifie cette génération. Dorénavant, il s'agit non plus seulement de corriger les erreurs du passé, mais de ne pas les répéter. Cette pandémie nous oblige à repenser l'université dans son ensemble et dans toute sa complexité. La crise a, certes, mis à nu des failles structurelles, mais elle ne les a pas créées. En ce sens, saisissons-nous de l'occasion pour les combler. L'urgence est absolue, et nous devons investir sur le long terme. Il faut, à mon sens, renforcer le principe d'autonomie des universités. Chaque composante présente une spécificité. et sportives (Staps). Ces particularités ne permettent pas aujourd'hui une application uniforme des mesures décidées par votre ministère. Il y a un vrai besoin de flexibilité Il faut de la cohérence, de la clarté et un cap. » Ce ne sont pas mes mots, madame la ministre ; ce sont ceux du chef de l'État. Les incessantes variations réglementaires constituent donc un défi. Pour ne plus courir de manière erratique après la crise, il faut cesser cette valse délétère de circulaires et présenter une stratégie de long terme. Il n'est plus possible qu'étudiants et enseignants aient pour seul gouvernail l'inconstance. Cette exigence est rendue encore plus urgente par la menace d'un nouveau confinement. Il faut aussi admettre que la formation des étudiants en ressort dégradée. Il est donc impératif d'y remédier. Pour cela, il faut non seulement préparer dès à présent la rentrée prochaine, mais aussi réfléchir à un plan de restructuration de l'enseignement supérieur. Pour terminer, l'effet de masse lié aux très bons résultats obtenus en licence amène à reconsidérer les modalités de sélection à l'entrée en master. Des pistes de réflexion existent. Les universitaires les tiennent à votre disposition. La crise sanitaire a le mérite de faire vaciller des certitudes établies, de questionner les discours dominants et de rappeler les décideurs à leur devoir d'humilité. Elle a vu aussi une remarquable mobilisation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour assurer au pied levé, dans des conditions difficiles, la continuité de leurs missions académiques. La France gagnerait à se réconcilier avec les acteurs de ses territoires en abandonnant ses tentations récurrentes de concentration, afin d'accepter de promouvoir une différenciation. Connaissance et reconnaissance vont de pair. C'est l'un des principaux défis des temps qui s'ouvrent. Le chantier est immense. Tout cela réclame ce qui a tant manqué jusqu'à présent : de l'anticipation, de la cohérence et des moyens à la hauteur de l'enjeu

Cette phrase-choc, rappelée par mon collègue et ami Pierre-Antoine Levi, devrait être complétée par : « On veut un vaccin, c'est plus sain ! » Il faut ouvrir au plus vite nos universités. Trop de destins, trop d'histoires, trop de vies, trop d'avenirs sont en jeu. Des artistes, des chercheurs, des entrepreneurs, des praticiens en herbe sont en pleine régression, en pause prolongée. sont en souffrance, beaucoup à l'agonie, en détresse, précarisés, hors sol, désorbités, sacrifiés. On préfère faire l'aumône d'un psy plutôt qu'offrir un vaccin. Demandez aux parents et aux grands-parents ce qu'ils pensent de cette catastrophe annoncée ! Il ne s'agit pas d'opposer une classe d'âge à une autre, une génération à une autre. Le serment d'Hippocrate ne fait pas de priorité entre un patient âgé et un jeune patient. Mais le serment d'Hippocrate constitue-t-il l'alpha et l'oméga de la conduite d'une nation ? Ne faut-il pas introduire un délit de non-assistance à génération en danger ? Surtout quand il faut compter sur elle pour prendre le relais, financer nos retraites, fonder des familles, inventer, créer et aller de l'avant Il n'y a pas que des décideurs politiques pour lancer l'idée d'une vaccination des étudiants comme prélude à la réouverture des universités et comme témoignage du prix que nous attachons à la jeunesse de notre pays. J'entends de grands médecins plaider pour une vaccination des étudiants. Le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, l'a proposée. Le professeur Jean-Luc Dumas, ancien doyen de la faculté de médecine de Bobigny, le rejoint. Cette stratégie de vaccination des étudiants est d'autant plus pertinente que le vaccin AstraZeneca ne semble pas adapté aux plus de 65 ans, comme le précisent les autorités de santé allemande et autrichienne. L'agence du médicament italienne recommande un « usage préférentiel » pour les 18-55 ans, et cette barre des 55 ans a également été retenue par le chef de l'unité de coordination anti-covid en Bulgarie. n'est pas contre-indiqué pour les plus de dix-huit ans. Bien au contraire : son taux de couverture est excellent ! Qui nous reprocherait de passer aux actes en faveur d'une vaccination étudiante ? Pas les 2,7 millions d'étudiants, ni leurs familles, ni la communauté pédagogique et encore moins le monde économique ! Mais qui demain ne nous le reprocherait pas si nous n'agissions pas aujourd'hui ?

Bien entendu, être vacciné ne signifie pas abandonner les gestes barrières individuels. Nous saurons le rappeler aux intéressés, et ils sauront prendre des engagements. Si le distanciel est devenu une modalité, voire une consigne, luttons de toutes nos forces pour que le présentiel demeure un acquis. C'est aussi la condition de la santé mentale de toute une génération en danger. La raison et la science nous permettent d'espérer. Il ne manque que le courage pour franchir le pas et, pour beaucoup, dont je suis, quitter cette zone d'inconfort qui consiste à laisser notre jeunesse dans les limbes, morts-vivants dans l'antichambre la vie ! La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le malaise grandissant des étudiants affectés par la crise covid inquiète. Leur précarité augmente massivement et accentue des situations déjà très fragiles. Les effets délétères de la situation et l'anxiété qu'elle suscite ont des conséquences graves sur la santé mentale des jeunes, accrues par l'isolement et les cours à distance. Décompensation, stress, dépression, idées de suicide ... les signaux de détresse et de souffrance psychologique sont multiples, même si les statistiques disponibles sont globalement insuffisantes. Les difficultés économiques sont provoquées en particulier par l'arrêt de nombreux jobs étudiants. Près de six sur dix ont réduit ou arrêté leur activité rémunérée en rendant leur location, entraînant ainsi l'arrêt de leurs études. Des demandes d'aide alimentaire les concernent massivement. Elles représentent à ce jour près de 30 % de l'augmentation. Certaines images de files d'attente ont légitimement choqué. L'aggravation de la situation s'observe également avec le sentiment d'une forme d'abandon et d'inutilité. S'estimant insuffisamment écoutés et sollicités par les pouvoirs publics, ces jeunes voient leur horizon s'obscurcir sans constater une réaction qui soit à leurs yeux à la hauteur des enjeux et de leur peur quant à l'avenir. Cette détérioration n'a été prise en compte que tardivement et de manière insuffisante, malgré de nombreuses alertes. Je mesure chaque jour la difficulté de la tâche du Gouvernement en cette période exceptionnelle. Mais nous devons tous ensemble être beaucoup plus exigeants en faveur du monde étudiant. en faveur du monde étudiant. Madame la ministre, tant que des mesures d'éradication du virus ne seront pas applicables, il faut de toute urgence adapter la stratégie du pays à tous les secteurs d'activité et n'abandonner personne. La vie sociale des jeunes étudiants est essentielle. Les dernières annonces du Gouvernement, bien que tardives, vont dans le bon sens, mais manquent d'ampleur : un jour par semaine en présentiel, avec une jauge maximale de 20 %, deux repas par jour à un euro, un accompagnement psychologique sous forme de chèque pour ceux qui sont en mal-être En tout cas, la toute récente décision qui leur permet de manger dans les espaces des Crous avec un protocole sanitaire renforcé va dans le bon sens et accompagne utilement le retour très partiel. Je tiens à vous remercier de votre engagement décisif en ce sens, madame la ministre. Je ne néglige pas d'autres aides décidées depuis le début de la crise, de la crise, parfois en décalage avec les ressentis de terrain et le vécu en temps réel des étudiants. J'ai eu copie de la lettre de la présidente de l'université de Franche-Comté et de Bourgogne, signée par d'autres présidents de composantes. Il y est fait référence à l'immense désespoir des étudiants, avec une interrogation

Donnez priorité aux échelons locaux de proximité les plus aptes à prendre en compte les difficultés sociales des étudiants. Régions, départements et villes ont un rôle plus important à jouer. Il faut leur garantir budgétairement les conditions d'une prise en charge optimale Aujourd'hui, c'est d'une dimension territoriale des solidarités dans la proximité que nous avons besoin. Des incompréhensions entre l'État et les territoires doivent être levées. Donnez Donnez priorité à un calendrier de reprise des cours en présentiel, en liaison avec une campagne volontariste de tests et de vaccination. Rien ne l'interdit à ce stade, malgré les incertitudes sur l'évolution de la pandémie. Cette génération est précieuse. Il faut que la vaccination soit effective pour toutes les étudiantes et tous les étudiants. Cela apportera la preuve de leur importance. Donnez priorité à l'action des collectivités locales pour accepter la mise en place des dispositifs d'emploi, de formation, de stages, adaptés à la période. Donnez priorité à chaque université, dans sa singularité et son autonomie, pour trouver des solutions appropriées à ses propres difficultés. L'institution elle-même a ses propres difficultés, mais elle est épuisée par les changements. Donnez priorité à la réflexion sur l'ensemble des dispositifs et critères d'aides, de bourses et de revenu étudiant de façon sérieuse, sans excès idéologique, mais sans tabou. Nous sommes pour une prise en compte améliorée des inégalités constatées ou vécues, sociales comme territoriales. Chaque étudiant doit pouvoir vivre dignement dans ses études, et non de ses études ! Les comparaisons internationales doivent nourrir utilement nos réflexions et inflexions. La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir organisé ce débat. Je suis très heureuse que la question des étudiants et de leur avenir intéresse la Haute Assemblée en ce début du mois de février 2021.

la question a été posée dès la sortie du premier confinement, avec une incertitude, qui ne vous aura pas échappé, sur les conditions sanitaires. Les établissements ont travaillé sur plusieurs scénarios. Ils ont travaillé sur une reprise en présentiel, que nous souhaitions tous ; elle a pu se faire, pour quelques semaines seulement malheureusement, puis elle a été en demi-jauge lorsque les cas de clusters ont commencé à apparaître dans les établissements, mais aussi lorsqu'un certain nombre de responsables politiques ont qualifié la situation dans les facultés de « catastrophique » et ont cru bon d'affirmer que la jeunesse accélérait la transmission du virus. J'ai toujours défendu le fait que les établissements d'enseignement supérieur n'étaient pas des lieux où l'on se contaminait en suivant les enseignements. Cela va me permettre de répondre à l'une de vos premières interrogations. Je pense que vous avez tous un jour ou l'autre fréquenté un campus universitaire.

pas. Avec les établissements, nous avons mis en place des protocoles pour trois étapes dès le début du mois de janvier.

au sein des écoles et des universités, ils n'avaient pas eu le temps de se faire des camarades. Certains d'entre eux venaient d'autres régions, voire d'autres pays.

ont évidemment été pris en charge, comme tout titulaire d'un contrat de travail. Tous ceux qui avaient des contrats d'apprentissage ont évidemment été accompagnés et aidés : si nous avons maintenu le nombre d'apprentis cette année, c'est parce que le Gouvernement a été présent auprès des entreprises pour faire en sorte que l'apprentissage ne soit pas sacrifié. Ceux qui avaient des contrats de professionnalisation ont pu les conserver.

Là encore, nous n'avons pas attendu pour agir. Dès le mois de juin, les loyers des résidences universitaires ont été gelés. Dès le mois de juin, nous avons annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation des frais d'inscription. Dès le mois de juin, nous avons, pour la deuxième année consécutive, augmenté les bourses sur critères sociaux. Nous avons

un mot sur l'accompagnement psychologique des étudiants. Nous avons mis en place différentes mesures sur le front de l'accompagnement humain.